La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

nous clôturons aujourd'hui près de quatre mois de travail sur un texte qui a presque quintuplé de volume et suscité de nombreux et intenses débats, que ce soit au Parlement ou dans la société civile. Je me réjouis que nous ayons pu aboutir à un accord avec nos collègues députés, même si, il faut le dire, ce n'est pas forcément le meilleur des deux textes, entre celui de l'Assemblée nationale et celui, plus ambitieux, du Sénat, qui a été finalement J'en prends pour exemple les mesures relatives à la régulation de la publicité et à la généralisation de l'affichage environnemental, pour lesquelles le Sénat avait développé une approche plus ambitieuse. Cela étant, nous revenons de loin, et ce texte permet de fixer un cap et d'envoyer un message clair pour engager durablement notre économie dans la transition bas-carbone, même si des mesures complémentaires seront nécessaires. Depuis le mouvement des « gilets jaunes » jusqu'à aujourd'hui, en passant par les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, nous avons affirmé une ambition environnementale à la hauteur des enjeux, à quelques mois de la COP26, et oeuvré dans le sens d'une réconciliation des transitions écologiques, économiques et sociales. Pour parvenir à un texte commun, nous avons tous, députés comme sénateurs, dû faire des compromis. Surtout, le plus important est assuré : les dispositions de ce texte vont entrer en vigueur rapidement. C'était impératif au regard de l'urgence climatique et de la nécessité d'accompagner nos concitoyens dans la transition écologique. Je pense que nous pouvons être satisfaits d'avoir ainsi agi en responsabilité. Heureusement, de nombreux apports du Sénat ont été préservés. Je pense à certaines mesures de régulation de la publicité, à la lutte contre l'écoblanchiment, au développement du vrac, au combat contre la prolifération des déchets dans la vente à emporter, aux mesures de facilitation de la rénovation et de la réparation des véhicules des particuliers et à la clarification juridique des atteintes les plus graves à l'environnement.

De votre côté, quel calendrier avez-vous défini pour la publication des très nombreux décrets d'application nécessaires pour préciser la mise en oeuvre de cette loi ? Pouvons-nous compter sur la célérité des administrations concernées pour « transformer l'essai » et préserver les équilibres que les parlementaires ont souhaité définir, entre accélération de la transition écologique et garantie de la justice sociale ? Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de revenir sur le détail du texte dans les prochains mois et années. Je répondrai évidemment : « Présente ! » La parole

mes chers collègues, Marta de Cidrac l'a dit, nous retrouver aujourd'hui ensemble pour adopter le texte de l'accord trouvé en commission mixte paritaire sur ce projet de loi aurait paru inespéré pour certains il y a quelques mois. Après avoir travaillé sur le fond des mesures qui nous étaient soumises, nous avions, au Sénat, retrouvé l'espoir d'aboutir à cet accord pour assurer l'essentiel : une entrée en vigueur rapide des mesures contenues dans ce texte. Les discussions dans les jours précédant la CMP et une certaine surenchère médiatique, à laquelle nous n'avons, nous, les rapporteurs, pas pris part, ont failli décevoir cet espoir. Mais nous y sommes arrivés, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis, car les compromis passés avec les députés dans le cadre de la CMP permettent au Sénat de préserver des mesures très importantes. Je pense aux avancées sur le verdissement et l'intégration de considérations sociales dans le droit de la commande publique. Je pense au volet agricole du projet de loi, dans lequel nous sommes parvenus à pousser des mesures qui engagent durablement notre agriculture dans la transition agroenvironnementale, tout en protégeant nos agriculteurs contre la concurrence déloyale. Je pense aux mesures innovantes que nous avons su préserver pour lutter contre la déforestation importée. Je pense, enfin, à la réforme du recul du trait de côte, pour laquelle nous avons garanti un partage des responsabilités entre l'État et les collectivités, partage qui devra être prolongé dans le cadre de l'examen du budget. J'ai, moi aussi, quelques regrets, sur la prise en compte insuffisante des activités humaines dans le cadre de la préservation des hydrosystèmes ou encore sur le refus du Gouvernement de prendre des mesures dédiées pour préserver notre souveraineté alimentaire. Sur le volet de la lutte contre la déforestation importée, nous aurions encore pu aller plus loin dans le pilotage des émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à ce phénomène. Même lorsque nous avions des désaccords avec les députés, nous avons cherché à trouver des solutions de compromis et à garantir la qualité et la clarté des normes qui s'imposeront demain à nos concitoyens et à nos entreprises. Il faut saluer cet exercice de démocratie parlementaire, dans lequel le Sénat montre, une fois de plus, qu'il ne dit jamais « non » par discipline ni « oui » par dogmatisme, mais qu'il est capable d'être force de propositions au service des grands enjeux de notre temps, au premier rang desquels figure la lutte contre le réchauffement climatique. Comme ma collègue Marta de Cidrac, je souhaite, madame la ministre, vous interroger sur la suite.

au moment du vote des conclusions de la commission mixte paritaire, je souhaite saluer le travail que nous avons su mener ensemble, loin des caricatures fausses et méprisantes à l'égard de la Haute Assemblée. Très bien il n'y a pas, au Sénat, de climatosceptiques ni de climato-inactifs, mais des acteurs d'une écologie pragmatique, d'une écologie de l'intelligence territoriale et d'une écologie de la vraie vie, qui ne porte pas les habits d'une loi-pénitence. J'en veux pour preuve les nombreuses avancées sénatoriales dans ce texte en matière de mobilité : moins de taxations, en évitant l'écotaxe sur l'ensemble du territoire, tout en réglant la question du sillon lorrain ; plus d'ambition, notamment sur le fret ferroviaire et fluvial plus d'accompagnement, avec le forfait mobilité durable rehaussé jusqu'à 600 euros et cumulable avec un abonnement de transport public ; la mesure prolongée de suramortissement pour nos poids lourds, pour répondre au réalisme du marché, en attendant la disponibilité des offres alternatives

ces travées, la baisse la TVA sur le train pour en faire un produit de première nécessité, n'a malheureusement pas été retenue. Pour autant, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons à la charge sur ce sujet, ... Très bien ! Exactement ! ... comme sur ceux de l'apprentissage gratuit et obligatoire du vélo, de la réduction des péages autoroutiers pour le covoiturage ou des services de location sociale pour les véhicules les moins polluants. Au moment de conclure, je souhaite remercier l'ensemble des rapporteurs, nos administrateurs et vous tous, mes chers collègues, du travail collectif accompli et du chemin parcouru en quelques mois. Je n'oublie pas les présidents Larcher, Retailleau et Longeot, pour leur écoute de chaque instant, et encore moins le de notre commission, Didier Mandelli. Cette loi Climat et résilience ne réglera pas, pas, tant s'en faut, la difficile question du réchauffement climatique, mais le Sénat a préparé le terrain pour que certains réveils soient plus ambitieux et moins douloureux. C'est avant tout une étape de concorde supplémentaire, qui enverra un message fort d'unité de la représentation nationale à nos concitoyens, au service d'une noble cause. La

par tous nos concitoyens, quelle que soit leur classe sociale. Le Sénat a obtenu des avancées significatives sur des points majeurs. Ainsi, alors que le texte était presque muet sur l'énergie, le Sénat a obtenu des avancées sur le nucléaire, sur l'hydroélectricité et sur l'hydrogène. Bravo ! Nous avons notamment obtenu la reconnaissance de la pertinence de l'énergie nucléaire dans l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050, ce qui n'était pas un petit combat. Nous sommes parvenus à un texte bien plus ambitieux, et d'ailleurs salué comme tel, en matière de rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi à une transition plus solidaire au bénéfice des plus modestes, avec un reste à charge minimal. Nous avons eu, tout au long de l'examen du texte, le souci d'associer les collectivités territoriales à cette transition,

Il y avait, madame la ministre, beaucoup de vents contraires qui allaient dans le sens d'un échec de cette CMP. Nous avons prouvé, ensemble, que le Sénat est en pointe sur le sujet du réchauffement climatique, s'attachant moins aux effets d'annonce qu'à l'efficacité réelle des mesures proposées.

partout en France, en métropole comme en outre-mer, nos concitoyens et nos territoires font face à la même urgence, celle d'une planète à bout de souffle, d'un climat qui se transforme en menace- malheureusement, nos voisins belges et allemands l'ont encore expérimenté récemment -et d'une biodiversité qui s'érode à une vitesse jamais vue depuis l'extinction des dinosaures. Oui, nous vivons des temps troublés et difficiles. Et si certains pouvaient croire qu'il n'y avait plus qu'à baisser les bras, aujourd'hui, avec cette loi, vous répondez très clairement que, non, notre avenir nous appartient.

Oui, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, un vent de changement souffle en France et dans le monde. Nous ne voulons plus continuer comme avant, enfermés dans un système absurde qui n'a à offrir que des inondations, des canicules et des tempêtes. Nous ne voulons plus poursuivre cette course folle vers l'abîme, avec son cortège de destruction et de souffrances. Il est de notre responsabilité- la vôtre et la mienne -d'agir pour sortir le pays de cette impasse et le placer droit vers l'avenir. notre responsabilité de construire dès aujourd'hui, dès maintenant, cette France résiliente, solidaire, juste et écologique que le pays attend. Et aujourd'hui, ici même, c'est cette responsabilité politique, morale et historique que nous prenons. Ce projet de loi est singulier à plus d'un titre. Tout d'abord, parce qu'il renoue un pacte de confiance avec les citoyennes et les citoyens de ce pays. Nous entendons trop souvent qu'ils ne sont plus intéressés par la, la que notre démocratie vacille inexorablement. Pourtant, 150 Françaises et Français ont répondu à l'appel du Président de la République. de métropole et d'outre-mer, agriculteurs, retraités, étudiants, cadres, infirmiers, venus de tous horizons et de tous les métiers, c'est une petite France qui s'est rassemblée pour travailler avec courage et détermination durant neuf mois. jaunes ? Cette Convention résonne bien au-delà de ce seul projet de loi et de ces seules mesures : elle montre que citoyenneté, engagement, esprit du service de tous ne sont pas des concepts du siècle dernier, mais des réalités bien vivantes. Elle montre que notre pays est riche de cette passion : la politique, dans ce qu'elle a de noble, de beau, de juste, l'envie de changer, de faire changer et d'inventer toujours un avenir meilleur pour soi et pour ses enfants. C'est aussi cela, la promesse républicaine. Je veux dire et redire à chacune et à chacun des 150 de la Convention que leur héritage est immense et qu'il ne se cantonne pas à ce texte,

En effet, et c'est l'ancienne députée qui vous parle, c'est bien du Parlement que naissent les grandes lois, ... Du Sénat ! ... celles qui ont changé le pays, celles qui ont accéléré les transformations tant attendues et tant espérées. Et aujourd'hui encore, la démocratie représentative montre sa force : le débat, les amendements, le travail législatif sont tout simplement le gage d'une démocratie qui existe, qui vit par l'engagement des élus de la Nation. Permettez-moi de saluer sincèrement le travail des rapporteurs, de mes collègues du Gouvernement et des groupes de la majorité et de l'opposition. Ensemble, malgré les divergences et les désaccords,

C'est une nécessité absolue, qui transcende les clivages et les appartenances. Si nous pouvons avoir des désaccords sur les moyens d'y parvenir, cette unité sur le but à atteindre est pour moi la promesse d'y arriver. La commission mixte paritaire s'est ainsi révélée conclusive. Je veux y voir la marque que nous pourrons tous ensemble réaliser la transition écologique et y associer l'ensemble des Françaises et des Français. C'est en tout cas l'ambition que je porte : réaliser les grandes transitions de notre temps avec toutes et tous. tous. Aujourd'hui, en votant ce texte, nous passons de 150 citoyens à 67 millions de Français. Nous engageons avec force la transformation de nos existences, de notre économie, de notre travail, de notre alimentation, de nos déplacements et de notre manière d'habiter la Terre.

c'est l'interdiction de l'écoblanchiment, ou encore une meilleure régulation de la publicité. Vous avez, à ce titre, souhaité l'instauration d'une première mesure d'interdiction des véhicules les plus polluants en 2028, madame la rapporteure Marta de Cidrac, et je m'en félicite. Voilà un aperçu de ce que nous offre le titre I de ce texte. engager la bascule culturelle ne suffit pas à changer de modèle. C'est nécessaire, impératif et incontournable, mais nous devons ici résoudre des problèmes majeurs, aujourd'hui, sans attendre que le changement infuse au long cours : il y a toute une économie à transformer, à décarboner ; il y a des emplois à créer ou à recréer dans nos territoires ; il y a des territoires qui n'attendent que de prendre le flambeau. C'est tout l'esprit du titre II inclure les causes environnementales et sociales dans les marchés publics, doter la France d'un modèle minier adapté à notre temps, décliner la programmation pluriannuelle de l'énergie dans les régions ... Ce sont autant d'avancées majeures, autant de victoires pour l'écologie que je porte. Je salue ici le travail réalisé avec les rapporteurs Anne-Catherine Loisier, Pascal Martin et Daniel Gremillet. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ce texte va aussi permettre de lutter, enfin, contre des situations qui sont une honte pour notre pays. Je pense tout d'abord aux 40 000 victimes annuelles de la pollution de l'air, aux dizaines de milliers de malades, aux familles endeuillées, aux vies bouleversées. Nous devons à chacune et à chacun un air pur. C'est aussi simple que cela. C'est cette responsabilité que nous prenons aujourd'hui avec le titre l'élargissement de la fin de vente des véhicules fossiles en 2040 aux poids lourds, aux autobus et aux autocars neufs ; l'accélération de la trajectoire de verdissement des flottes d'entreprises, des collectivités et de l'État

Par ailleurs, monsieur le rapporteur Philippe Tabarot, comme vous l'avez souhaité, nous allons expérimenter le prêt à taux zéro pour déterminer son efficacité et renforcer le forfait mobilité durable. Mettre un terme à des situations honteuses, c'est aussi mettre un terme aux passoires thermiques injustes socialement, économiquement et climatiquement : 2 millions de Français grelottent l'hiver, transpirent l'été payent des factures exorbitantes, tout cela en émettant du CO2 que nous pourrions éviter. Grâce au travail parlementaire, ce texte pose une trajectoire d'interdiction de la mise en location. Il pose le cadre d'un changement durable et effectif et d'une véritable transformation. Ne nous leurrons pas : c'est un effort réel que nous demandons à des milliers de propriétaires, qui doivent pouvoir compter sur la solidarité de la Nation et sur le soutien de l'État. Je pense tout d'abord aux « accompagnateurs rénovation » : partout dans les territoires, ils viendront à la rencontre des Français pour les aider dans leur projet- choix de l'artisan, planning des travaux ... -, et cela du Ce soutien, c'est aussi le prêt « avance mutation », qui permettra de faciliter, pour des milliers de propriétaires, le financement des travaux. Ce soutien, enfin, je ne puis l'imaginer que dans la durée, car ce grand chantier de la rénovation s'étend bien au-delà de nos mandats. Pour réussir, nous devons donner aux Français de la prévisibilité et de la confiance dans le soutien public. Ils n'en ont pas avec vous ! Avec ce texte, nous gravons dans le marbre un principe d'engagement de l'État, qui garantira à nos concitoyens, notamment les plus modestes, un reste à charge faible. Je salue ici le travail du rapporteur Dominique Estrosi Sassone, qui a contribué à clarifier et à muscler la définition d'une rénovation performante. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, cette transformation dont je vous parle, c'est aussi celle du bon sens. Le bon sens qui consiste à ne pas construire de centres commerciaux au milieu des champs. Le bon sens qui consiste à cesser d'artificialiser contre nature, d'étendre nos villes, de fabriquer de l'isolement social et du sentiment d'oubli, en ravageant la biodiversité. Oui, nous allons diviser le rythme d'artificialisation d'ici à 2030. C'est un défi majeur pour les collectivités locales, et je salue le travail mené ici avec le rapporteur Jean-Baptiste Blanc. Telle est la portée du titre IV, qui transforme nos habitats et nos manières de vivre sur la terre en tournant la page d'un temps absurde et injuste.

un menu végétarien hebdomadaire dans les écoles et une option végétarienne quotidienne dans les universités. Des écoliers aux étudiants, tous nos jeunes auront accès à des menus savoureux et équilibrés, quel que soit leur régime alimentaire.

J'éprouve une fierté particulière à la lecture du titre VII, en ce qu'il porte la marque de notre apprentissage démocratique au long cours, en ce qu'il traduit notre responsabilité, bien au-delà de nos mandats, en nous dotant d'une gouvernance climatique à même de veiller à l'application effective de ce texte.

issu de cette volonté de changement, de cet esprit de transformation qui a façonné notre histoire. Il est issu d'heures de travail de citoyens, mais aussi de parlementaires, et issu d'une commission mixte paritaire que tous- moi la première -, annonçaient comme impossible. Pourtant, vous l'avez fait

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

Nous nous félicitons particulièrement des échanges qui ont eu lieu au Sénat. Ils ont permis de rappeler, si besoin était, que la Haute Assemblée est ancrée dans la réalité et déploie des solutions concrètes afin de répondre aux besoins des citoyens. Territoires s'est attaché, dès le début, à faire en sorte que ce texte ne vienne pas accentuer les fractures entre nos territoires. Nous l'avons dit, les solutions doivent être territorialisées pour être efficaces et acceptables. Nous le répétons, nous vivons un moment particulier dans la crise que nous traversons. Notre force sera d'utiliser la relance, afin d'accélérer notre transition écologique. Celle-ci doit être juste économiquement et socialement, respecter un calendrier précis. Elle doit surtout être efficace aux yeux des Français. et Territoires continue son combat et ses efforts pour une écologie libérale et humaniste, loin des incantations à la décroissance. La préservation de l'environnement et le soutien à la transition énergétique sont dans l'ADN de notre groupe. Pour nous, les solutions se nomment innovation, recherche et développement, financements verts, entreprises innovantes et progrès. Bref, comme l'a justement déclaré Bill Gates, nous avons besoin d'une transformation technologique sans précédent pour réaliser cette transition. Notre lutte contre le dérèglement climatique ne s'intensifiera que si nous décarbonons des pans entiers, fortement émetteurs, de notre industrie, que si l'énergie que nous consommons et produisons est propre, grâce à des innovations, tant dans le nucléaire que dans le renouvelable. Ainsi, nous regrettons que certains sujets fondamentaux, autour desquels nous allons devoir développer une réflexion et une action, n'aient pas été évoqués ou l'aient été La publication, le 14 juillet dernier, par la Commission européenne, de douze propositions de textes afin d'ajuster l'Union à son objectif de 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon de 2030 est pleine d'enseignements. Si les discussions seront longues et difficiles et que les promulgations de textes ne sont pas attendues avant 2023, les lignes sont plus claires, et le paquet beaucoup plus ambitieux que ce sur quoi nous avons pu nous entendre dans ce projet de loi. L'incitation est de mise et le coeur du problème est évoqué. Nous avons eu l'occasion de le dire, nombre de réponses émaneront des échelles européenne et mondiale. Notre projet de loi, nous le déplorons, privilégie un mode plus punitif.

Cependant, des avancées importantes, sur de nombreux sujets, sont au rendez-vous dans ces 350 articles. Je pense notamment au code minier, à la protection équilibrée des écosystèmes et de la biodiversité, aux certificats de production de biogaz,

Le travail est pourtant loin d'être terminé. Comme vous l'avez souligné, madame la ministre, plus une semaine ne passe sans qu'une catastrophe naturelle, à l'image des inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique, et en Belgique, nous rappelle l'urgence climatique dans laquelle nous nous trouvons et ses impacts dévastateurs sur nos populations. Nous sommes désormais tous conscients de l'enjeu immense qui se dresse devant nous et devant les générations futures. Nous serons au rendez-vous, mais il faudra aller beaucoup plus loin que ce projet de loi. Nos efforts sont désormais tournés vers Bruxelles. Espérons que la présidence française du Conseil de l'Union européenne soit à la hauteur de ces enjeux. La parole

nous le savons tous, aux enjeux quantitatifs de réduction d'émissions de CO2 qu'exige la communauté scientifique. Lundi dernier, sénatrices, sénateurs, députées et députés ont donc trouvé un accord en commission mixte paritaire.

les rapporteurs pour leur important travail, dans un temps très court. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts et sont restés attentifs aux propositions des différents groupes du Sénat ; qu'ils en soient remerciés. Toutefois, ce travail parlementaire montre que la recherche de compromis nous amène à des mesures, quantitativement totalement insuffisantes. Or justement, de manière quasi unanime, le Sénat avait tenu à inscrire dans le premier article de ce texte, qui a survécu à la paritaire, le respect de l'objectif européen de réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et sa déclinaison française. Nous connaissons depuis quelques jours la proposition de la Commission européenne pour la France

Il nous faudra donc, dans les toutes prochaines années, rehausser fortement notre ambition et voter de nouvelles mesures à fort impact carbone. Nous aurons alors, sans nul doute, à nous replonger dans les propositions de la Convention citoyenne.

propositions étaient assez modérées au regard de certaines des mesures proposées aujourd'hui par la Commission européenne, comme la fin des véhicules thermiques en 2035 ou l'objectif de production de 40 % d'énergie dès 2030 à partir de sources renouvelables,

lors de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, à adopter un autre texte, « raccord » avec le cadre européen. Le débat ne fait donc que s'ouvrir.

nous devions donc de crédibiliser, par nos propres mesures, l'engagement européen, seul levier susceptible d'entraîner, avant la COP de Glasgow, une dynamique pour un effort mondial équitablement réparti et à la hauteur de l'enjeu. Cette loi ne répond pas à cette urgence, raison pour laquelle le groupe écologiste n'a d'autre choix que de voter contre les conclusions de cette commission mixte paritaire.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « l'essentiel est de posséder une forte volonté et la persévérance », disait le grand poète allemand Goethe. De la volonté et de la persévérance, nous en avons eu, le 12 juillet dernier, près de neuf heures durant. Je veux ici, au nom de mon groupe, saluer le formidable esprit constructif qui a notamment animé nos deux présidents de commission, ainsi que nos rapporteurs. Sans eux et sans leur farouche volonté d'aboutir à une commission mixte paritaire conclusive, rien n'aurait été rendu possible. Le Sénat a fait oeuvre utile, et nous avons su collectivement, malgré toutes nos différences, nous montrer à la hauteur de l'enjeu qui se trouve devant nous. Je le dis d'autant plus facilement que nous n'étions pas forcément en phase, les uns et les autres, sur toutes les options défendues par notre assemblée sénatoriale, mais que nous étions animés d'une seule et même volonté aboutir et donner tout son sens à cette transition écologique que nous appelons de nos voeux et qui s'incarne dans ce texte issu d'échanges nourris et d'un très important travail entre les rapporteurs de nos chambres.

Madame la ministre, le bicamérisme a été au rendez-vous de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est une victoire qui n'a pas de prix, surtout sur un texte aussi essentiel, auquel d'aucuns prédisaient une issue défavorable. Nous avons su faire mentir pronostics et autres sondages, qui, sous couvert d'un climatoscepticisme sénatorial, donnaient peu de chances d'aboutir à nos travaux. Pourtant, sur des sujets aussi divers que les transports, l'énergie, la publicité, l'artificialisation des sols, le logement, les engrais azotés, la notion d'écocide,

Relever le défi de la transition écologique engage notre responsabilité : celle d'additionner les volontés de toutes et de tous, non d'exclure ni de diviser. Nous en avons donné l'exemple. J'espère que cela permettra d'entraîner tous nos concitoyens, partout sur le territoire, dans cette belle aventure de la transition écologique. Non, cette loi n'est pas une loi des petits pas, comme certains la caricaturent. Les faits sont têtus : cette loi est une contribution engagée et engageante au respect des accords de Paris de 2015, à l'agenda 2030 des objectifs de développement durable ou encore au Pacte vert pour l'Europe.

et son cumul avec un abonnement de transport en commun ; ensuite, cette mesure emblématique, dont nous ne partagions pas tous la substantifique moelle, défendue avec force et conviction par notre collègue Philippe Tabarot, sur le prêt à taux zéro dans le cadre de la mise en oeuvre des zones à faibles émissions. Oui, mes chers collègues, la transformation écologique passera avant tout par un changement des comportements. Et ce changement, c'est maintenant, pour reprendre un slogan qui a fait florès voilà quelques années. Assumons collectivement le fait de privilégier l'information des consommateurs et les incitations, plutôt que les interdictions arbitraires, souvent teintées d'anticapitalisme primaire. J'ai souvent dit, et je le répète une fois encore, l'écologie partagée, c'est celle qui tend vers l'idéal, mais qui comprend le réel. Ce texte nous aidera à tenir nos engagements climatiques : il contribuera à amplifier la transformation écologique de la société et à orienter notre économie vers la décarbonation. Économie, justice sociale et écologie sont compatibles, nous ne cessons d'oeuvrer à leur conjugaison. La vie d'un parlementaire est jalonnée de succès et d'échecs, mais rien ne peut remplacer ce sentiment d'avoir fait oeuvre utile et de contribuer, même très modestement, à une aventure collective et entraînante dont nous pourrons, dès demain, mesurer les effets. C'est le cas avec cette dernière étape et ce beau vainqueur qu'est, n'en déplaise aux contempteurs de tous poils et de tous bords, la transition écologique partagée par toutes et tous. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera bien évidemment ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, grâce au Sénat, ce projet de loi a pu être habité de l'esprit de justice sociale qui devait l'animer dès le départ, conformément à la mission attribuée à la Convention citoyenne pour le climat. Il revient désormais au Gouvernement, qui dispose dans notre pays d'un pouvoir budgétaire presque absolu, de renforcer cet aspect essentiel, pour accélérer la lutte contre le dérèglement climatique. Sans ce paramètre, faute d'accompagnement social et d'adhésion de nos concitoyens, toute transition vers un modèle économique et sociétal écologiquement plus vertueux sera vouée à l'échec. Aussi, il était légitime que le Sénat ne cède pas sur la création d'un prêt à taux zéro pour l'acquisition de véhicules légers. La mise en place de zones à faibles émissions mobilité discriminera une partie de nos concitoyens, qui, rappelons-le, se déplacent en premier lieu pour se rendre au travail. Le recours à la voiture ne constitue pas toujours une solution de confort, en raison d'une offre de transports qui ne répond pas aux besoins exprimés en termes de régularité, de fréquence ou encore d'accessibilité pour tous. Tant que le prix des véhicules électriques ou à hydrogène restera élevé et que les bornes électriques ou les points d'avitaillement en hydrogène ne seront pas aisément accessibles, la bascule vers les mobilités propres ne s'opérera pas. Par ailleurs, les reculs de la commission mixte paritaire quant à la TVA à 5,5 % pour les billets de train et l'instauration d'un dispositif de fixation d'un prix plancher pour certains billets d'avion sont incompréhensibles. L'examen du projet de loi au Sénat a également permis de doter ce texte d'un véritable volet consacré à l'énergie. Aussi, les dispositions relatives au développement de l'hydrogène ou encore favorisant l'hydroélectricité sont bienvenues. Cependant, je me réjouis de la suppression par la commission mixte paritaire des entraves au développement de l'éolien par le Sénat. Dans un tout autre domaine, je considère que la réforme du droit pénal de l'environnement méritait bien mieux : le recours à une circonstance aggravante en matière d'atteintes graves à l'environnement, plutôt que la création d'un délit générique sanctionnant l'ensemble des atteintes à l'environnement, est regrettable. Mes chers collègues, je tiens à saluer le travail accompli pour que la commission mixte paritaire puisse aboutir à un accord si inattendu. La tâche était délicate, mais la volonté des parlementaires était au rendez-vous pour tenter de préserver les progrès apportés par chacune des deux chambres par rapport au texte initial. Malheureusement, le résultat final demeure quelque peu décevant au regard de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre que nous nous sommes fixé pour 2030, relevé de 40 % à 55 % par la Commission européenne, qui a présenté, la semaine dernière, une série de mesures ambitieuses. Nombreux sont ceux qui dénoncent une loi frappée d'obsolescence avant même sa promulgation. Si elle intervient effectivement dans tous les domaines de la vie des Français, comme ne cesse de le rappeler le Gouvernement, ces changements seront imperceptibles face à l'ampleur des effets du réchauffement climatique. Les délais d'application de nombreux articles demeurent fixés à une échéance bien trop lointaine. C'est notamment le cas en matière de rénovation énergétique. Et ce n'est pas la possibilité pour le bailleur de donner congé au locataire pour réaliser les travaux, introduite par le Sénat et que je perçois comme dangereuse, qui changera la donne. Ainsi, chaque année perdue signifie que, à l'avenir, les efforts devront être multipliés dans un laps de temps plus serré, au risque d'alimenter les résistances sociales. Le projet de loi contient toutefois un certain nombre d'avancées qui ont le mérite d'exister, par lesquelles il est procédé à des ajustements nécessaires de notre politique environnementale : affichage environnemental, encadrement de la publicité et des allégations environnementales, développement du vrac, verdissement de la commande publique, réforme du code minier, lutte contre l'artificialisation des sols, malgré l'absence de mesures véritablement efficaces pour protéger les terres agricoles ... Pour toutes ces raisons, la majorité de mon groupe s'abstiendra. La parole est à Mme Marie-Claude

à l'issue de longues heures de discussion en séance publique, puis en commission mixte paritaire, le Parlement aura abouti à un texte commun. Loin du satisfecit que s'est accordé à lui-même le Gouvernement, nous gardons un goût amer de l'examen de ce projet de loi. Je tiens néanmoins à souligner la qualité du travail mené en commission, notamment de la part de nos rapporteurs. Que dire des 300 articles qui constituent ce texte, si ce n'est que, malgré quelques avancées, ils sont un empilement de mesures anecdotiques de loi extrêmement bavard traduit une politique des petits pas qui n'est pas à la hauteur des changements économiques et sociaux imposés par la crise écologique. Les associations environnementales et les 150 citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi le Conseil économique, social et environnemental et le Haut Conseil pour le climat, tous déplorent le manque d'ambition de ce texte. Alors que l'Union européenne, en lançant son plan pour atteindre une baisse de 55 % des émissions à l'horizon 2030, montre une certaine volonté, même s'il y aurait à y redire, la France reste à la traîne, y compris dans les échanges avec ses homologues européens. Le Conseil d'État vient pourtant de nous ordonner de prendre d'ici à neuf mois des mesures concrètes pour le climat, dans le cadre de « l'affaire du siècle ». Mes chers collègues, il y a urgence, et même urgence absolue

Exodes, phénomènes climatiques extrêmes, malnutrition, extinction d'espèces ... La vie sur terre sera inéluctablement transformée bien avant 2050. Le rapport se conclut ainsi : « Nous avons besoin d'une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. » La gestion des irrecevabilités a d'ailleurs bien confirmé cette absence de volonté de s'attaquer à des sujets de fond, comme le rééquilibrage des pouvoirs et la redistribution des richesses, exclus de la discussion. mobiliser de nouvelles ressources et des moyens humains supplémentaires pour construire un projet de développement au bénéfice d'un avenir durable rendant la transition socialement acceptable n'est pas à l'ordre du jour : pas de plan de financement à la hauteur pour le rail, pas de taxe sur les transactions financières, pas de taxe sur les dividendes, pas d'écocontribution sur les billets d'avion, aucune taxe sur les surfaces commerciales qui participent à l'artificialisation des sols et toujours aucune conditionnalité des aides publiques. Alors que le Sénat avait introduit un taux de TVA à 5,5 % sur les billets de train, la CMP est revenue sur cette avancée initialement proposée par la Convention citoyenne. Les entreprises publiques, dans des secteurs aussi importants que les transports et l'énergie, sont exclues des débats, alors qu'elles constituent, il faut bien le dire, des leviers évidents pour accompagner cette politique de transition écologique. J'en veux pour preuve le projet Hercule, qui procède du démantèlement d'EDF. Quant aux enjeux de l'habitat, ils sont sous-évalués, l'obligation de rénovation thermique ne concernant qu'une infime partie du parc et l'interdiction de la location de passoires thermiques étant reportée à 2028. Cet exercice législatif est une opération de communication destinée à verdir la politique gouvernementale en cette période préélectorale. Il ne répondra pas aux enjeux climatiques, car la feuille de route confirmée par le Président de la République reste la même, faisant prévaloir les intérêts financiers privés sur l'intérêt général, le temps court du profit sur le temps long de l'intérêt commun. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, après une commission mixte paritaire historiquement longue, nous achevons aujourd'hui l'examen de ce projet de loi qui aurait dû être une étape cruciale dans la conversion de notre pays à une écologie du quotidien. J'ai eu la chance de participer à ce petit cénacle, davantage en position de spectateur, je dois le dire, qu'en tant que véritable participant. À chaque point dur abordé, une suspension de séance, des arbitrages en attente de Matignon ; les tractations allèrent ainsi bon train à l'abri des oppositions. L'acmé de cette séquence fut sûrement la discussion sur le prêt à taux zéro pour l'achat d'un véhicule peu polluant, que nous avions ici même adopté quasi unanimement. Nous avons tenu bon face aux arguments abscons du rapporteur Cazeneuve et des députés La République En Marche. Ceux-ci défendaient un dispositif de microcrédit

sur le taux de TVA à 5,5 % pour les billets de train, qui ne figure plus dans le texte final. Comment pouvons-nous favoriser le report modal de nos déplacements si nous ne rendons pas attractifs les trajets ferroviaires ? Nous sommes donc en présence d'un texte le plus petit dénominateur commun entre l'Assemblée nationale et le Sénat ; ainsi pouvons-nous précisément évaluer l'ambition écologique de cette loi, qu'il faut mettre en regard de nos objectifs climatiques et des propositions initiales de la Convention citoyenne pour le climat. Au risque de faire figure de trouble-fête des majorités sénatoriale et gouvernementale, cette loi n'atteint pas les objectifs que nous nous étions assignés. De l'aveu même de Pascal Canfin, une nouvelle loi devra être proposée dès 2022. Nous ne sommes donc pas dans les clous de la trajectoire bas-carbone fixée par l'accord de Paris. Nous n'avons pas le temps de revenir point par point sur chaque titre pour mesurer l'étendue de nos déceptions quant à cette loi souvent plus bavarde que véritablement opérante. Quelques exemples, néanmoins, pour vous en convaincre, mes chers collègues. Tout d'abord, à l'article 1, le Sénat et l'Assemblée nationale ont réussi l'exploit de créer un affichage environnemental invisible, puisqu'il sera seulement accessible sur internet. Quel décalage avec notre réalité climatique, devenue, elle, bien visible ! De surcroît, tous nos efforts pour intégrer des critères sociaux ont été balayés. L'expérimentation est élargie à cinq ans au lieu de dix-huit mois. Seul le textile sera finalement concerné par une obligation d'affichage. Nous sommes là bien en retrait de la loi anti-gaspillage et pour une La mise en place d'un Éco-score ou d'un « score carbone », dont vous vous targuez, madame la ministre, est réduite à une coquille vide pour laquelle aucun cadre précis n'est établi et qui ne permettra qu'à la marge d'améliorer l'information du consommateur. Le travail de sape dirigé contre la proposition de la Convention citoyenne a fait son oeuvre. envisageable de conserver la mention du niveau de rémunération des agriculteurs dans l'affichage environnemental. Mais non ! Le Gouvernement préfère créer, dans la loi Égalim 2, un « Rémunéra-score » ... On empile les labels, les scores, au lieu de proposer un affichage unique, clair et utile aux Français.

Enfin, nous avons assisté à la suppression de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles de notre collègue Nicole Bonnefoy, que nous avions eu la sagesse d'intégrer au présent projet de loi. Selon le rapporteur Cazeneuve, il faut se garder de préempter l'examen de la proposition de loi copiée-collée par un député de La République En Marche ! Les inondations cataclysmiques qui frappent nos voisins belges et allemands nous invitent en effet à attendre plutôt qu'à anticiper est des mesures tendant à lutter contre la pollution des sols, mesures promues par notre collègue Gisèle Jourda. Comparé à l'ambition initiale de la Convention citoyenne pour le climat, ce texte de loi peine à traduire le message d'urgence écologique que les 150 nous ont transmis.

en bout de course d'un quinquennat manqué pour la transition écologique et solidaire : rien sur l'écoresponsabilité des entreprises, rien sur la résilience de notre modèle économique face au changement climatique, trop peu sur l'accompagnement social ou sur le développement du fret ferroviaire, ce dernier étant pourtant indispensable à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre l'écocide, il est travesti en délit ... Nous avions besoin d'une loi-cadre ; vous nous proposez un catalogue de mesures disparates dont nous devrons attendre les décrets d'application.

Mais nous en sommes trop loin, et le paquet européen adopté mercredi dernier nous le rappelle puissamment. Ainsi voterons-nous contre ce texte. Il n'offre que trop peu d'outils pour lutter efficacement contre l'insécurité écologique qui sera demain notre quotidien. La parole est

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, autant le dire d'emblée : que la CMP sur le projet de loi Climat et résilience ait abouti est pour nous une immense satisfaction. Nous n'étions pas nombreux à y croire. Et pour cause : la tâche était colossale et le terrain miné. Comment négocier, en quelques jours seulement, 377 articles tous plus sensibles les uns que les autres ? Le Gouvernement nous y a aidés en acceptant que la date de cette CMP soit quelque peu repoussée, afin, donc, de nous laisser un peu de temps pour travailler- je vous en remercie, Malgré ce délai supplémentaire, le pari n'était pas gagné d'avance, comme en témoigne la longueur historique de cette commission mixte paritaire : neuf heures de débat-

de conserver les apports et les acquis du Sénat. De fait, nous en avons conservé beaucoup : sur les 311 articles restant dans le texte établi par la CMP, 103 proviennent du Sénat ; nous pouvons collectivement nous en féliciter. en féliciter. Toutefois, l'actif du Sénat ne doit pas seulement être analysé de façon quantitative : il doit l'être aussi d'un point de vue qualitatif, car nous avons rehaussé l'ambition environnementale de ce projet de loi.

Surtout, nous avons supprimé un angle mort, avec la prise en compte du nucléaire comme atout nécessaire pour décarboner notre mix énergétique et accompagner l'essor des énergies renouvelables. Enfin, nous avons introduit des mesures relatives à la forêt- cet égard le travail d'Anne-Catherine Loisier -, en renforçant son rôle stratégique de puits de carbone ou en définissant un objectif de préservation de la qualité des sols forestiers. Pour relever le défi climatique, le « défi du siècle », comme certains l'appellent, il nous faut être bien plus ambitieux que nous ne l'avons été jusqu'ici. Mais l'expérience prouve aussi que l'on ne mènera pas une transition environnementale digne de ce nom sans qu'elle soit acceptée par nos concitoyens et déclinée sur le terrain. C'est cette idée forte qui a structuré nos travaux : il n'y aura pas de transition environnementale sans justice sociale et sans mobilisation territoriale, de justice sociale, c'est toujours s'interroger sur l'acceptabilité des mesures prises. Or nombreux sont nos concitoyens à fustiger « l'écologie punitive Vous n'aimez pas ce terme, madame la ministre, mais c'est une réalité qu'il désigne. Il faut réconcilier les Français avec l'écologie. C'est selon nous la seule manière de ne pas opposer transition écologique et économie de montrer que la première peut aussi être porteuse de croissance, d'innovations, de bien-être et d'emploi, à condition de créer l'écosystème économique, si vous me passez l'expression, qui le permette.

En outre, je le disais, il n'est pas de transition écologique sans mobilisation territoriale. C'est pourquoi nous regrettons la suppression de l'article 1 A, qui donnait, enfin, aux collectivités les moyens

est aussi l'esprit de la disposition que nous avons adoptée concernant les écotaxes régionales. Je suis satisfait d'un compromis qui permet, sur l'initiative de notre assemblée, de conserver une approche différenciée et pragmatique en restreignant la mesure aux régions frontalières. Il s'agit en effet de répondre à un réel enjeu, à savoir le report de trafic étranger, tout en évitant un dispositif qui affecterait de manière disproportionnée des régions qui n'en auraient ni l'utilité ni la volonté L'ambition environnementale est donc concrétisée par un souci de justice sociale et de mobilisation territoriale. Mais,, rien ne se fera sans l'Europe. Et il ne vous étonnera guère, mes chers collègues, qu'un centriste conclue par un mot européen. Tout ce que nous avons fait ici s'inscrit dans un cadre communautaire, et même mondial, celui d'engagements climatiques que nous devons respecter. Tel est le sens de l'article 1 AA, adopté à l'unanimité de notre assemblée : rappeler que la France doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre en se conformant aux objectifs de l'Union européenne et de l'accord de Paris, des objectifs transnationaux dont la France a été l'un des principaux artisans. Or, en avril dernier, l'Union européenne a revu à la hausse les ambitions européennes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Le texte que mon groupe s'apprête à voter

que la Commission vient de présenter, c'est-à-dire d'imposer le nouvel objectif communautaire à tous nos partenaires. Il serait impensable qu'elle ne s'y conforme pas elle-même dans le même temps. Très bien

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je souhaite en cet instant avoir une pensée pour les victimes du drame qui s'est déroulé chez nos voisins allemands et belges la semaine dernière. Le bilan est lourd, dramatique même : 191 personnes décédées et plus d'une centaine de disparus. Au moment où je vous parle, l'ouest des États-Unis est ravagé par de terribles incendies. En une journée, hier, dans l'Oregon, ce ne sont pas moins de 1 200 kilomètres carrés qui ont été réduits en fumée, et actuellement des milliers de personnes sont évacuées. puissance et leur soudaineté, font écho à celles que nous avons nous-mêmes vécues très récemment dans le sud de la France- la tempête Alex. Nous subissons aujourd'hui les conséquences d'un dérèglement climatique qui ne connaît évidemment pas de frontières.

Nous avions tant entendu parler de sa préparation la Convention citoyenne pour le climat et les différentes déclarations du Président de la République et des membres du Gouvernement que nous avons été déçus de découvrir un projet de loi dont la portée normative était relativement réduite : des mesures symboliques, ne permettant pas d'endiguer le réchauffement climatique et de traiter l'ensemble de ses conséquences. En examinant ce texte, nous ne nous sommes pas demandé comment être plus verts ou plus réalistes ; nous avons souhaité que le Sénat contribue à la politique publique environnementale en restant fidèle à sa tradition, c'est-à-dire en échappant aux affrontements stériles entre défenseurs à tout prix de l'environnement et défenseurs de l'économie.

en un mot des femmes et des hommes responsables. Nous avons commencé ces débats animés par un objectif commun : permettre à la France de répondre à ces défis majeurs. J'en veux pour preuve l'article additionnel avant l'article 1,

défendre les positions du Sénat, bien sûr, qui permettent d'aller plus loin sur de nombreux sujets, prendre en considération cette urgence climatique et la nécessité de mettre en oeuvre très rapidement les mesures Après neuf heures de négociations difficiles avec nos collègues de l'Assemblée nationale, nous sommes finalement parvenus à un accord en commission mixte paritaire, et ce, je tiens à le dire, malgré l'attitude parfois détestable du rapporteur général de la Je dois le reconnaître, cet accord était pour le moins inespéré, tant les sujets de divergence entre le Sénat et l'Assemblée étaient nombreux. Je souhaite en cet instant remercier tout particulièrement nos collègues membres de la CMP, les rapporteurs, bien sûr, et nos équipes d'administrateurs,

quelques chiffres, tout d'abord, pour illustrer les résultats de ces négociations : sur les 377 articles examinés, 111 conservent la rédaction du Sénat, 158 sont le fruit d'une rédaction de compromis. Ces négociations ont donc permis de conserver de nombreuses mesures très fortes introduites par le Sénat. Ainsi, le prêt à taux zéro destiné à accompagner les ménages les plus modestes dans le renouvellement de leurs véhicules a été conservé, après presque une heure d'interruption de séance. Il s'agit d'une mesure de bon sens : personne ne

La CMP a également conservé les apports du Sénat quant à la nécessité de rendre la commande publique plus exemplaire, avec l'intégration de considérations sociales et la prise en compte des objectifs de développement durable.

De même, la CMP a maintenu dans le texte l'ajout du Sénat concernant la possibilité pour les communes situées sur le littoral d'installer des centrales solaires sur les sites dégradés. Cette modification significative du droit résulte d'un travail de longue haleine et répond à une demande répétée des collectivités du littoral. Les précédents intervenants ont détaillé la plupart des mesures, sur lesquelles je ne reviendrai donc pas plus avant. Bien entendu, nous avons dû faire des concessions- je pense notamment à la TVA à

Nous devons continuer à agir, en tant que parlementaires, bien sûr, en tant que citoyens, en tant que consommateurs, à tous les niveaux, pour apporter la plus forte contribution possible à l'atteinte des objectifs définis. Il n'y a pas, madame la ministre, mes chers collègues, de gagnants ni de perdants là où il s'agit du climat et de l'avenir de nos enfants. Ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, ni votre ministère, ni le Gouvernement ne sortent vainqueurs de ce marathon législatif. Il reste beaucoup à faire,

à la pertinence de toutes les décisions ou positions que vous pourrez prendre sur les sujets qui touchent au quotidien de nos concitoyens. Le groupe Les Républicains votera majoritairement ce texte.

Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements précédemment adoptés par le Sénat,

La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents, réunie ce jour, sont consultables sur le site du Sénat. En l'absence d'observations, je les considère comme adoptées.- L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,chacun le sait, la politique de développement solidaire est le complément indispensable de notre action diplomatique et militaire. Elle répond à la fois à une exigence de justice et à une logique d'influence, tout en étant indispensable pour notre propre prospérité et sécurité à long terme- ce doit être gagnant-gagnant. Je salue donc le travail accompli par les deux assemblées pour améliorer ce projet de loi ; il a permis de préciser de nombreux points et de combler des lacunes. En particulier, le Sénat a renforcé la transparence de la politique de développement solidaire, en complétant les informations devant figurer dans le rapport global prévu à l'article 2, qui devra faire l'objet d'un débat dans les deux assemblées. Par ailleurs, le texte adopté en commission mixte paritaire permettra aussi- et c'est un autre apport du Sénat

essentiellement par le biais de dons et de prêts très concessionnels ; d'autre part, le financement, principalement par des prêts non concessionnels, des biens publics mondiaux et de la convergence économique dans les pays à revenu intermédiaire. Il nous semblait important

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui à l'issue de la commission mixte paritaire du 24 juin dernier, longtemps attendu, constitue une avancée importante pour notre politique de solidarité internationale. Le passage au Parlement a en effet permis de concrétiser le travail accompli depuis plusieurs années par les commissions des affaires étrangères des deux assemblées. Il traduit également votre engagement, monsieur le ministre, à mener à son terme un processus long et semé d'embûches, dont la crise sanitaire n'a pas été la moindre. Ce projet de loi fixe ainsi un cadre clair et précis pour l'ensemble des principes et des finalités de cette politique de solidarité internationale. À cet égard, l'ajout d'un article liminaire résumant ses grands axes constitue un apport pertinent des députés, dont nous avons souhaité renforcer encore la portée, en distinguant trois aspects principaux la lutte contre la pauvreté et les inégalités internationales ; la préservation des biens publics mondiaux ; la défense des droits humains. Chacun de ces grands objectifs, d'égale importance, doit se déployer selon une logique qui lui est propre, avec des instruments financiers spécifiques. L'intelligibilité de la loi et l'adhésion de nos concitoyens à cette politique souvent très méconnue supposaient cette clarification, que les députés ont pleinement approuvée. Nous nous félicitons également des dispositions améliorant la gouvernance de l'aide publique au développement, même si nous aurions souhaité aller plus loin dans ce domaine. Le texte introduit certes un peu plus de cohérence, mais nous estimons que le rôle de chef d'orchestre du ministre chargé du développement devrait davantage être affirmé, notamment en ce qui concerne le pilotage de l'Agence française de développement. S'agissant des dispositions financières, nous avions, dès le début de l'examen du texte, relevé le paradoxe que constituait une loi de programmation qui ne prévoyait pas de crédits au-delà de 2022. Loi de programmation rétrospective », « loi dont les objectifs sont atteints avant même d'être votés » : les qualificatifs quelque peu ironiques, mais malheureusement assez fondés, n'ont pas manqué, aussi bien de notre part que de celle des députés. Au Sénat, nous avions tenté d'y remédier par l'introduction d'une programmation des crédits de la mission « Aide publique au développement » jusqu'en 2025. Les députés, tout en voulant maintenir un objectif de 0,7 % du RNB en 2025, s'y sont opposés. Finalement, nous nous sommes accordés sur une trajectoire de croissance avec des pourcentages du RNB pour chaque année jusqu'en 2025. Il s'agit maintenant de traduire cette trajectoire au sein des lois de finances successives afin de donner à cette politique les moyens de ses ambitions. La commission mixte paritaire a également permis d'aboutir à un accord sur un autre aspect très novateur du texte : la création d'une commission d'évaluation de l'aide publique au développement, sujet sur lequel le président de notre commission, Christian Cambon, s'est particulièrement engagé. Nous avions ici une différence d'appréciation notable avec les députés qui souhaitaient, sur le modèle britannique, une commission purement administrative et technique avec des experts à temps plein. Nous estimions de notre côté qu'une commission équilibrée devait comporter parmi ses membres des parlementaires, capables d'apporter un regard différent, soucieux de l'efficacité concrète des projets et motivés par le contrôle démocratique de cette politique. Nous avons trouvé un accord combinant les deux approches, en prévoyant au sein de la même commission un groupe d'experts indépendants rendant compte de ses travaux à un collège de parlementaires. Cette commission permettra ainsi de mesurer l'impact final des projets et d'apporter de nombreuses informations à l'Assemblée nationale et au Sénat afin que le Parlement puisse exercer le rôle de contrôle de l'action du Gouvernement qui lui est confié par la Constitution. Par ailleurs, nous avons également trouvé un accord avec les députés s'agissant des dispositions relatives au ciblage de l'aide, que nous avions introduites lors de l'examen du texte par notre commission. C'est la première fois qu'est ainsi fixé dans la loi un triple objectif : part comparée des dons et des prêts ; part des crédits bilatéraux par rapport aux crédits multilatéraux ; concentration sur les pays prioritaires. Je rappelle que ceux-ci sont les pays africains les plus en difficulté, notamment les pays du Sahel, ainsi qu'Haïti, dont il est inutile de rappeler la situation critique. En fixant ainsi de véritables obligations de résultat pour la concentration des moyens sur les pays qui en ont le plus besoin, nous tenons, me semble-t-il, une véritable avancée. Celle-ci prend tout son sens au moment où la réduction du format de nos forces engagées au Sahel a été annoncée par le Président de la République. On le sait, le développement de cette région est la condition de sa stabilité à long terme et nous devons être plus que jamais aux côtés des États concernés pour soutenir tous les efforts qu'ils entreprendront au bénéfice de leurs populations.

mois, est essentiel pour l'avenir de notre diplomatie, dont le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales constituent désormais l'un des piliers, alors que la vie internationale est marquée par d'immenses défis, à commencer par la pandémie et l'urgence environnementale. Chacun le sait désormais, ces défis qui ont partout de très graves conséquences appellent des solutions collectives, qui doivent aussi s'inventer au Sud. C'est le sens de ce projet de loi auquel l'Assemblée nationale, puis le Sénat ont manifesté leur soutien. Les deux chambres ont apporté de précieux enrichissements, que les travaux de la commission mixte paritaire du 24 juin ont permis de concilier. Le texte renforcé et équilibré qui en résulte reçoit le plein accord du Gouvernement. Nous avons proposé un texte d'ambition qui dote notre politique de développement solidaire de moyens fortement accrus. Nous avons proposé un texte pragmatique qui définit des géographies et des enjeux prioritaires en parfaite cohérence avec les engagements politiques de la France. Nous avons proposé un texte à la fois stratégique et humaniste, c'est-à-dire porteur d'une véritable géopolitique des valeurs françaises, mais aussi européennes. Nous avons présenté ce texte pour proposer à nos partenaires du Sud une autre voie que celle de la dépendance, voire de la sujétion à des acteurs qui ne cherchent qu'à étendre leur emprise. leur emprise. Il s'agit de les accompagner sur la voie d'une souveraineté renforcée, préoccupation que nous partageons pleinement et que nous mettons également en oeuvre pour nous-mêmes au sein de l'Union européenne. Nous avons proposé ce texte pour construire sur la scène internationale un autre chemin que celui de la brutalisation et du « chacun pour soi », qui ne peut mener qu'à un échec collectif. Souvent, au-delà des clivages politiques, nos débats l'ont montré, la représentation nationale s'est reconnue dans ces grandes orientations. Mieux, vous avez eu à coeur de les décliner de manière encore plus précise, tout en faisant droit aux contraintes avec lesquelles nous devons tous composer, si nous voulons agir et construire une véritable différence. Je veux aujourd'hui saluer à la fois l'esprit d'exigence et de responsabilité, dont vous avez fait preuve, et le dialogue constant, constructif et fructueux que nous avons mené ensemble tout au long de ces mois de travail. Notre réussite, je tiens à le redire cet après-midi, doit aussi beaucoup à l'engagement ancien et permanent du président Cambon de la regrettée Marielle de Sarnez, dont le président Bourlanges poursuit aujourd'hui les efforts. Ce travail doit aussi beaucoup à Hervé Berville, à Hugues Saury et à Rachid Temal, qui ont oeuvré ensemble, jusque dans la dernière ligne droite, pour que nous aboutissions à ce résultat dont nous pouvons collectivement être fiers. Je tiens aussi à remercier devant vous Jean-Baptiste Lemoyne, qui m'a accompagné avec beaucoup d'efficacité tout au long de l'examen de ce projet de loi devant le Parlement. Le Gouvernement se réjouit que vous soyez parvenus à un accord avec l'Assemblée nationale sur l'article 1 qui fixe les moyens consacrés à l'aide publique au développement. La rédaction retenue réaffirme notre volonté collective de concrétiser l'engagement du Président de la République de consacrer 0,55 % de la richesse nationale à notre aide publique

trajectoire jusqu'en 2025 et la difficulté de prévoir des chiffres en valeur absolue, notamment du fait de l'évolution de la part non pilotable de notre aide publique au développement. Je sais que votre assemblée tenait à ce que soit inscrite une trajectoire des moyens accordés à l'aide publique au développement jusqu'en 2025. La rédaction retenue est un bon compromis qui permet de répondre en grande partie à cette préoccupation, puisque le texte prévoit, au-delà des crédits budgétaires pour l'année 2022, des cibles intermédiaires à titre indicatif en pourcentage du RNB pour les années 2023 et 2024. comme le Gouvernement s'y était engagé, le texte prévoit que la représentation nationale sera consultée sur la programmation des crédits avant la fin de l'année 2022. Nous partageons par ailleurs avec vous- je sais que vous y êtes particulièrement attachés -la volonté de concentrer notre aide sur les pays les plus vulnérables, en particulier Nous avons eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises lors des débats sur les projets de loi de finances successifs et dans le cadre de l'examen de ce projet de loi. Des propositions en ce sens ont été faites par votre assemblée pour mieux cibler notre aide publique au développement. de la flexibilité introduite par le texte issu de la commission mixte paritaire, qui permettra de concilier nos différents objectifs : concentration de la composante bilatérale de l'APD,

Ainsi, ce texte permet de définir des priorités claires sur les canaux, les instruments et les pays prioritaires, tout en mettant en place les éléments de souplesse nécessaires. Cet équilibre,

Cette concentration de nos efforts va de pair avec la logique partenariale de notre politique de développement. On ne saurait concevoir le développement aujourd'hui comme on le pratiquait hier. Il s'agit de faire davantage avec nos partenaires, et pas simplement pour eux. On ne le répétera jamais assez : imposer des solutions de l'extérieur à nos partenaires du Sud serait aussi politiquement critiquable que pratiquement inefficace. Nous faisons de plus en plus face à des défis communs ; c'est donc forcément ensemble que nous devons inventer les solutions pour y répondre.

qui mettent en oeuvre cette politique est également essentielle à son efficacité, car ces acteurs agissent le plus souvent au plus près des populations. Je tiens également, parmi les avancées permises par vos travaux, à souligner la création d'un dispositif de restitution des produits de cession des biens dits mal acquis introduit par l'Assemblée nationale. Il a fait l'objet d'un large consensus au sein des différents groupes politiques. Je veux ici rendre hommage à Jean-Pierre Sueur : son implication et les propositions qu'il a formulées sur ce sujet ont été décisives. Ce dispositif constitue un moyen très concret de lutter contre les ravages de la corruption et de la prévarication. À ce titre, il s'inscrit parfaitement dans l'esprit de notre texte. Des précisions tout à fait bienvenues ont été apportées au cours des débats au Sénat. Je me félicite de la formulation de compromis adoptée par la commission mixte paritaire, qui garantit la compatibilité de ce dispositif avec nos obligations découlant de la convention des Nations unies contre la corruption, en permettant aux populations concernées de bénéficier des richesses dont elles ont été spoliées. Le Gouvernement se réjouit, en outre, des dispositions introduites sur l'initiative de vos rapporteurs pour mieux définir et encadrer l'action de l'Agence française de développement, qui contribue à la mise en oeuvre de la politique de développement définie par l'État, et les missions de service public exercées par Expertise France. Le texte prévoit très clairement un renforcement du pilotage par l'État de notre politique de développement. C'était une forte demande de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il était nécessaire que ce projet de loi y réponde : cela nous permettra de mieux garantir que les actions que nous menons et que nous finançons correspondent aux objectifs stratégiques que nous nous sommes fixés. La chaîne de décision et de gouvernance est ainsi clarifiée du plus haut niveau, avec le Conseil présidentiel du développement, en passant par nos opérateurs, notamment l'Agence française de développement, jusque dans nos pays partenaires où le rôle dévolu aux ambassadrices et aux ambassadeurs sera renforcé dans le cadre d'un conseil local du développement qui rassemblera régulièrement, sous leur présidence, toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette politique au quotidien, en lien direct avec les populations bénéficiaires.

Au-delà des modes de désignation des personnalités qualifiées, qui seront précisés par décret, il est essentiel de veiller à ce que les membres de cette commission ne reçoivent pas d'instructions, ne subissent pas de pressions et disposent d'un mandat dont la durée soit suffisamment longue pour leur permettre de travailler sereinement, en présence de parlementaires. Ces conditions sont désormais réunies. Le Gouvernement, je le dis en particulier au président Cambon qui est très attaché à ce sujet, est déterminé à ce que cette commission d'évaluation indépendante voie le jour le plus rapidement possible. La hausse des moyens engagés depuis le début du quinquennat rend nécessaire de renforcer encore davantage ce que les instances internationales de développement Je me félicite également que la commission mixte paritaire ait trouvé un accord sur le nouveau dispositif d'attractivité des organisations internationales prévu dans ce projet de loi. Comme vous le savez, le Gouvernement est très attaché à ce dispositif qui, sans méconnaître les droits du Parlement, doit permettre de renforcer notre activité internationale. l'enjeu est de placer notre pays au centre du combat pour le développement et les biens publics mondiaux. Nous devons en effet chercher à conjuguer influence et attractivité dans un contexte où la diplomatie des biens communs s'inscrit désormais dans un ensemble de dynamiques aussi géopolitiques que d'autres sujets. Ce dispositif nous permettra d'aller plus vite dès le début, puisqu'il ne sera plus nécessaire d'attendre la loi autorisant la ratification de l'accord de siège. Les privilèges et immunités pourront être octroyés immédiatement, mais le Parlement sera amené à se prononcer trois fois : d'abord sur l'habilitation, puis sur la ratification de l'ordonnance et, enfin, sur l'autorisation de ratification de l'accord de siège. Je tiens aussi à vous remercier d'avoir enrichi notre cadre de partenariat global. Ce document est d'une importance majeure dans la mesure où il expose à l'intention de nos partenaires, comme d'ailleurs de nos concitoyens, la philosophie qui préside au renouveau de notre politique de développement, ses grandes priorités géographiques et sectorielles, ainsi que son architecture de pilotage et sa trajectoire globale. Il propose également un cadre qui permettra de mesurer les résultats atteints dans les pays partenaires

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, protéger vraiment la France, les Françaises et les Français des bouleversements, des instabilités et des crises internationales suppose de construire avec nos partenaires du Sud la voie d'un développement qui

C'était l'occasion pour nous d'exprimer toutes nos attentes autour de ce pilier, encore si fragile, de la politique étrangère française. Car cette aide n'est pas facultative, elle n'est pas un geste de charité : c'est une responsabilité.

Nous n'avons pas, loin de là, réussi à éradiquer la faim dans le monde : aujourd'hui, ce sont encore 690 millions d'êtres humains, soit 10 % de l'humanité, qui souffrent de la faim. Ce chiffre est en augmentation à cause de la crise climatique, tout comme celui de l'extrême pauvreté.

Le rôle des organisations de la société civile est formellement reconnu- cela a été rappelé -et les financements qui transitent par elles sont voués à augmenter. L'égalité des genres est enfin consacrée comme une priorité transversale, une place accrue est accordée à la jeunesse et les peuples autochtones sont pris en compte. Le groupe écologiste, qui défendait tous ces points et bien d'autres, tient à saluer les améliorations apportées par le Sénat. Nous voterons donc majoritairement en faveur de ce projet de loi, bien que les conclusions de la commission mixte paritaire se soient traduites par des reculs regrettables. Ces reculs portent d'abord sur des demandes des ONG

budgétaire est atrophiée. L'objectif de 0,7 % reste mollement inscrit, mais cette programmation n'est fixée en valeur absolue que jusqu'à l'année prochaine, et non plus, comme nous l'avions proposé, jusqu'en 2025. ces conditions de loi de programmation ? Ce manque de visibilité est particulièrement dommageable pour nos partenaires, en particulier les ONG. Enfin, la trajectoire budgétaire en hausse, en quelque sorte esquissée au crayon à papier, ne peut endiguer la montée des inégalités mondiales que si elle s'accompagne d'une lutte contre les causes de ces inégalités, aux premiers rangs desquelles un modèle économique qui n'est favorable ni aux populations ni à l'environnement. Sans cette dimension, l'APD demeure, je l'ai déjà dit, le pansement sur la jambe de bois du système capitaliste. La vision que nous portons en tant qu'écologistes est celle d'une APD libérée des logiques de rentabilité et des impératifs de la diplomatie économique française. Nous regrettons profondément de n'avoir pu infléchir le texte en ce sens.

également comme objectif l'exigence d'une transparence et d'une responsabilité accrues pour tous les organismes qui contribuent à notre influence à l'étranger. Enfin, le dépassement des logiques de rentabilité aurait dû nous permettre de consacrer davantage aux pays les plus pauvres, ce qui devrait être le premier but de notre APD. Le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires continuera de porter ces objectifs qui sont les seuls à même de faire de l'aide au développement un véritable pilier de notre politique extérieure.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de notre réunion d'aujourd'hui sur les conclusions de la Cette séance marque l'achèvement d'un long processus législatif entamé en 2018. Je tiens à remercier tout d'abord le président de notre commission et les deux rapporteurs, ainsi que le rapporteur de l'Assemblée nationale. Je salue leur état d'esprit constructif. Le chemin a été long et semé d'embûches, mais grâce à votre détermination, monsieur le ministre, le cap a été maintenu.

La semaine dernière, cinq agences de l'ONU ont publié des données qui montrent combien il est urgent de renforcer notre mobilisation pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Face à cette urgence, nous avions le devoir de nous entendre sur un de nous entendre sur un texte de compromis. L'objectif fixé par le Gouvernement est atteint. Le texte que nous nous apprêtons à adopter confère un

et plus durables. En bonne intelligence, nous avons réussi à dépasser nos divergences qui, bien que peu nombreuses, concernaient des dispositions majeures. Pour la première fois, le Gouvernement a eu le courage de proposer l'inscription dans la loi d'une véritable programmation budgétaire pour notre APD. Le texte établi par la commission mixte paritaire prévoit une programmation ambitieuse et réaliste.

figurent dans le texte : la remise d'une lettre annuelle d'objectifs au directeur de l'AFD ; le rôle central joué par les collectivités d'outre-mer et par les organisations de la société civile, ce qui n'est pas évident pour un vieux pays colbertiste comme le nôtre

que, en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je me réjouisse du renforcement des compétences des conseillers des Français de l'étranger, qui seront membres de droit des conseils locaux de développement.

si la crise sanitaire n'en finit pas de questionner nos systèmes économiques et sociaux, elle a aussi permis de souligner avec force le caractère incontournable de notre politique de développement. Annoncé depuis 2018 et repoussé à plusieurs reprises, l'examen de ce projet de loi de programmation était un rendez-vous législatif très attendu. L'objectif du texte est de fixer le cap de notre politique de développement pour les prochaines années. En effet, après les orientations définies par le comité interministériel de la coopération internationale et du développement (Cicid) au début du quinquennat, notamment l'objectif d'atteindre un niveau ambitieux d'aide publique au développement de 0,55 % du RNB en 2022,

Toutefois, ce retard est largement imputable à la crise sanitaire, dont les conséquences économiques et sociales ont bousculé le cours de nos travaux ces derniers mois. Cela étant dit, je salue le travail de longue haleine des rapporteurs, nos collègues Hugues Saury et Rachid Temal, du président Christian Cambon, ainsi que du rapporteur pour avis de la commission des finances, le président de notre groupe, Leurs travaux ont permis, en premier lieu, de faire converger les positions des commissions des affaires étrangères et des finances au sein de notre assemblée et, en second lieu, de parvenir à un accord lors de la commission mixte paritaire. Le texte élaboré par celle-ci conserve un nombre significatif d'apports du Sénat, témoignant de l'esprit constructif qui a animé nos débats. À ce titre, l'accord trouvé sur la programmation définie à l'article 1 constitue une évolution majeure par rapport à la proposition initiale du Gouvernement. Je tiens à rappeler le constat unanime selon lequel l'intérêt budgétaire de ce texte était initialement très limité, puisque l'article 1 se contentait essentiellement d'entériner les moyens budgétaires déjà validés par le Parlement. Afin d'adopter une réelle loi de programmation, le Sénat avait, en première lecture, prolongé la trajectoire des crédits de la mission jusqu'en 2025, avec une clause de revoyure à mi-parcours. Si la commission mixte paritaire n'a pas retenu cette trajectoire des crédits de paiement, elle a en revanche conforté le caractère programmatique de ce projet de loi, en proposant une trajectoire exprimée en pourcentage du RNB jusqu'en 2025. Nous pouvons nous réjouir de cet accord qui permet de préserver l'effort budgétaire de la France en matière de développement pour les prochaines années. Quant à la part de taxe sur les transactions financières (TTF) affectée au développement, le plafond actuel a été sanctuarisé et il nous reviendra de conduire un nouveau débat sur cette question lors de l'examen du prochain projet de loi de finances. Un accord a également été trouvé sur d'autres apports du Sénat, tels que les objectifs chiffrés pour la part de l'aide publique bilatérale, pour la composante dons et pour l'aide pays programmable. Les précisions apportées par le Sénat sur la restitution des biens mal acquis ont également été préservées, tout comme les dispositions relatives à l'information du Parlement, notamment aux articles 2 et 10 . Je souhaiterais terminer en saluant l'accord trouvé sur les dispositions relatives à la commission d'évaluation de l'aide publique au développement, placée auprès de la Cour des comptes. Une meilleure évaluation de l'efficacité de cette politique est nécessaire dans un contexte de croissance de ses moyens budgétaires, alors que nos finances publiques connaissent de fortes contraintes. La définition de cette nouvelle instance, inspirée de l'exemple britannique, a nourri des débats animés au sein de notre assemblée. L'équilibre que nous avons trouvé contribue à améliorer la transparence de la politique de développement, tout en préservant le rôle constitutionnel d'évaluation alloué au Parlement. Enfin, il témoigne, s'il fallait encore en apporter la preuve, de la qualité de l'intérêt du travail parlementaire pour enrichir et préciser les textes qui nous sont soumis. Nous sommes donc bien sûr favorables à ce texte. La parole

qui visait à programmer, enfin, un effort d'APD digne d'un pays comme la France, et la faiblesse des engagements concrets qu'il contenait. Après le passage en commission mixte paritaire, rien ne s'est amélioré de ce point de vue, bien au contraire

Mais aucun engagement réellement précis ne permet de garantir la trajectoire. Tout reste hypothétique et ce texte n'est toujours pas une loi de programmation. Surtout si on le compare à la loi de programmation militaire, comparaison pertinente, puisque le Gouvernement prétend viser l'équilibre au sein du triptyque des 3D- diplomatie, défense, développement. D'un côté, la loi de programmation militaire comprend des engagements financiers d'ampleur pour faire ou préparer la guerre ; de l'autre, l'APD est toujours beaucoup trop faible pour lutter contre les inégalités mondiales-

paritaire, les quelques ajouts du Sénat ont été réduits comme peau de chagrin. La programmation budgétaire n'a de programmation que le nom, comme je viens de le dire. Nous allons voter en vérité, pour l'essentiel, une loi de finances anticipée sur une ligne budgétaire réduite à l'année 2022. La formulation très hypothétique de cet article montre l'absence de volonté budgétaire réelle du Gouvernement. Alors que le Sénat avait adopté

Autre enjeu de nos batailles lors des débats de mai dernier, la question des cibles de l'APD. Nous avons, assez collectivement, partagé un constat : notre APD était jusqu'ici trop orientée vers les prêts et peu accessible aux pays qui

bien éloigné du nécessaire contrôle politique. C'est en tout cas ce que nous craignons. Au terme de cette navette parlementaire, il reste le sentiment que la France rate le coche et qu'elle ne se donne pas, une fois de plus, les moyens ambitieux dont elle proclame Pourtant, tout, de la pandémie à l'échec de l'opération Barkhane, nous appelle à réviser nos concepts de coopération pour passer de la protection de nos intérêts de puissance à une véritable stratégie de développement pour tous les peuples, centrée sur la maîtrise par les pays visés par l'APD des moyens de leur développement et par la mobilisation de leurs ressources internes, parmi lesquelles figurent notamment les instruments monétaires et fiscaux. De ce point de vue, il est significatif que tous les amendements que nous avons proposés visant à des réorientations structurelles, par exemple sur les recettes fiscales des pays pauvres de droits de tirage spéciaux (DTS), comme cela vient d'ailleurs d'être décidé pour le Liban, aient été rejetés. Au-delà de l'insuffisance de nos engagements budgétaires, c'est le sens même de notre politique de développement qui reste problématique. Nous maintenons notre abstention

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'accord trouvé entre les députés et les sénateurs en commission mixte paritaire sur le projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités aboutit à un texte transpartisan. Ce texte concrétise de nouvelles ambitions pour notre politique de développement solidaire. Il vise à être un levier puissant de la diplomatie et du rayonnement de notre pays. Il ouvre la voie à une stratégie claire et à des priorités fonctionnelles et géographiques. Les actions d'aide publique au développement menées pourront également bénéficier d'un réel dispositif d'évaluation. Je souhaite, à cette occasion, remercier nos collègues de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, notamment nos rapporteurs Hugues Saury et Rachid Temal et bien évidemment notre président Christian Cambon, pour leurs travaux et leur écoute tout au long de l'examen de ce texte. Dans le cadre de mon mandat de représentant des Français établis hors de France, et à la faveur de mes multiples déplacements en circonscription, j'ai pu constater sur le terrain l'importance vitale de notre aide publique au développement et de son opérateur, l'Agence française de développement. J'espère que l'aboutissement de ce projet de loi suscitera une nouvelle impulsion afin que l'aide soit allouée de manière efficace aux pays qui en ont le plus besoin. Le texte comprend désormais une programmation financière solide, quelle que soit l'évolution de notre PIB. Une clause de revoyure est prévue une consultation et un vote du Parlement avant la fin de 2022 pour les trois années suivantes l'objectif est d'atteindre 0,7 % du RNB en 2025, comme vous l'avez dit, monsieur le ministre, conformément aux engagements pris par la France devant les Nations unies. La part de la taxe sur les transactions financières versée au Fonds de solidarité pour le développement ne pourra pas être inférieure à 528 millions d'euros. Ce fonds devra financer des biens publics mondiaux, comme la santé, l'éducation et la lutte contre le changement climatique. Dans un délai de six mois, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport portant sur l'amélioration de l'utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières. La commission d'évaluation de l'aide publique au développement, créée à l'article 9 du projet de loi, préserve le rôle de contrôle de nos deux assemblées. Le texte présente une définition plus claire des cibles pour la composition de l'aide au développement, entre l'aide bilatérale et l'aide multilatérale, entre les prêts et les dons, entre les pays à revenus intermédiaires et les pays pauvres prioritaires. Un équilibre entre un certain fléchage et le besoin de souplesse a été trouvé : la composante bilatérale de l'aide publique au développement devra atteindre en moyenne 65 % du total de l'aide sur la période 2022-2025 les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l'aide. Nous nous réjouissons que de nombreux apports du groupe Union Centriste aient été conservés à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire. La reconnaissance de nos territoires d'outre-mer comme véritables atouts stratégiques et les politiques en faveur des droits des enfants complètent le texte présenté aujourd'hui. permettront de favoriser l'apprentissage du français et la francophonie, outils indispensables de notre rayonnement à l'international. À titre personnel, je me réjouis que mes deux amendements aient prospéré à l'issue de la

dispositions qu'elles permettent aux TPE-PME de droit local détenues par des entrepreneurs français à l'étranger de bénéficier d'un accès facilité au crédit, par le biais de garanties offertes par l'AFD. Comme j'ai eu l'opportunité de l'exprimer à de nombreuses reprises dans cet hémicycle, cette solution financière est souhaitée depuis de nombreuses années afin de permettre à ces entrepreneurs de contribuer au développement des pays qui les accueillent. Les entrepreneurs français à l'étranger sont des vecteurs de l'efficacité de notre politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales : ils méritent tout notre soutien. Mes chers collègues, ce texte sur l'aide publique au développement est ambitieux. Il reflète une certaine idée française de la solidarité, pour reprendre votre belle formule, monsieur le ministre.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons place une fois de plus sous nos yeux, avec un « effet loupe », les inégalités de ce monde. L'accès aux vaccins et aux soins est très inégal. Or la lutte contre la pandémie doit se faire à l'échelle planétaire : notre situation dépend grandement de celle des autres parties du monde. aussi le cas pour les inégalités mondiales, qui sont encore plus profondes, et cet exemple doit nous convaincre d'accentuer encore nos efforts. Appréhender notre rôle nous renforce dans la conviction que, dans un monde toujours plus interconnecté, l'aide publique au développement est essentielle et doit être mieux dirigée. Rappelons-nous que cette aide est aussi dans notre intérêt, condition pour bâtir des équilibres à la fois mondiaux et internes. Le groupe Les Indépendants se félicite de l'issue conclusive de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi. Les deux assemblées ont travaillé étroitement afin de trouver un consensus qui nous incite à une action réfléchie et plus efficace. Ainsi, la fixation du niveau de dépenses, accompagnée de dates, est un bon moyen d'atteindre les objectifs financiers d'aide au développement que nous nous sommes donnés.

D'autres limites sont aussi inscrites dans le « dur » de la loi : je pense notamment à la limite basse du produit de taxe sur les transactions financières affecté au Fonds de solidarité pour le développement. La boussole de ce texte est l'efficacité de notre aide, à la fois en termes de pilotage, avec des objectifs clarifiés en matière de programmation, et de soutien. En effet, la redirection de l'aide publique au développement vers les pays les plus prioritaires était nécessaire. La prise en compte des indicateurs du programme de développement durable l'était tout autant. De la même manière, une composante bilatérale de l'aide fixée à 65 % est un signe positif, tout comme sa traduction en une part importante de dons.

Enfin, et notre groupe tenait particulièrement à ce point, nous saluons la place renforcée de la société civile dans notre aide publique au développement. La société civile est en effet, monsieur le ministre, un véritable compas pour orienter l'aide au développement en fonction des besoins des populations dans les pays destinataires,

L'aide publique au développement, son orientation, son niveau, ses priorités, son efficacité devaient être réformés. C'est chose faite. C'est pourquoi le groupe Les Indépendants votera en faveur de l'adoption des conclusions de cette commission mixte paritaire. Notre pays est l'un des plus grands contributeurs mondiaux de l'aide au développement. Le travail et les efforts que la France y consacre et doit continuer à y consacrer ne seront pas suffisants, si le reste du monde n'ajoute pas sa pierre à l'édifice. Nous devrons donc poursuivre nos actions

Nous avons travaillé rigoureusement, avec une grande exigence et la volonté de faire aboutir une loi sur l'aide publique au développement qui n'avait que trop tardé. Avec nos collègues de l'Assemblée nationale, nous sommes parvenus, je le pense, à un bon compromis. Je voudrais féliciter les corapporteurs, Hugues Saury et Rachid Temal, qui ont pu, tout au long de nos débats, bénéficier du soutien de la très large majorité du Sénat et, bien sûr, du groupe socialiste. Grâce à ces travaux, notre assemblée s'est illustrée par des avancées notoires. Nous avons rétabli une trajectoire financière qui n'apparaît plus du tout tronquée, comme c'était le cas dans le projet de loi initial. Nous allons voter des engagements chiffrés, malheureusement en pourcentage seulement, mais jusqu'en 2025, date à laquelle nous devrons atteindre les 0,7 % du RNB-

Il nous faudra cependant être particulièrement vigilants, car derrière un affichage qui peut paraître ambitieux aujourd'hui les engagements réels et concrets sont ténus. Parce qu'il nous est apparu que l'aide française souffrait d'une forte dispersion, ce qui ne favorise pas son efficacité, nous avons souhaité la cibler mieux, comme l'ont dit

Enfin, ce texte comprend des avancées sur l'ensemble des questions de genre et sur une meilleure prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Je dois souligner le rôle très important joué par la délégation aux droits des femmes du Sénat à cet égard. Nous nous félicitons aussi que la France s'engage à promouvoir les principes de la convention lutte contre les violences faites aux filles et aux femmes. Tout au long de nos débats, nous avons été, d'une certaine façon, des lanceurs d'alerte, que ce soit sur la levée des brevets, sur les vaccins ou sur la constitution d'états civils fiables, autant de sujets que le Gouvernement n'a pas voulu prendre en compte dans le texte, mais qui sont désormais sur la table des négociations. La pandémie nécessite des réponses mondiales. Alors que nous avons en France- croyez-moi ! -des débats de riches, les populations des pays pauvres attendent de pouvoir se faire vacciner et ainsi de sauver leur vie. Enfin, permettez-moi de lister tout ce qui manque, de mon point de vue, dans ce texte, des points sur lesquels les socialistes vont continuer de se battre pour faire bouger les lignes. Vous avez mis un terme à l'ambition de cibler 60 % de la taxe sur les transactions financières vers le Fonds de solidarité cette taxe atteint aujourd'hui des montants records : elle a rapporté plus de 1,7 milliard d'euros en 2020, elle aurait donc permis d'alimenter de façon considérable les ressources affectées à l'aide au développement. Dans six mois, lors de la remise du rapport qui

à l'égard de tous les acteurs, publics et privés, qui exercent une influence à l'étranger afin de prévenir, de dénoncer et de sanctionner des atteintes portées aux droits humains, aux libertés fondamentales

que le principe de non-discrimination fait partie des piliers de l'État de droit. Ce principe a été récemment réaffirmé par le Président de la République lors de la conférence nationale humanitaire, mais vous ne l'avez pas traduit dans le texte et il reste extrêmement flou. L'article 13 du présent projet de loi fait référence à un rapport qui va affiner la doctrine française en la matière. Il devrait nous être présenté prochainement- nous l'attendons. Nous attendons aussi que le Gouvernement s'engage pour sécuriser l'action de l'ensemble des organisations internationales humanitaires, particulièrement dans les zones de conflit et de crise, comme au Sahel. Mes chers collègues, vous le voyez, pour nous, beaucoup de combats restent encore à mener, mais ce texte permet des avancées qui seront utiles aux acteurs de l'aide publique au développement. Par conséquent, les socialistes le voteront. le voteront. Ce sera pour nous un geste de fraternité en direction des populations les plus pauvres du monde. La

collègues, nous y voilà enfin : nous sommes arrivés au terme d'un long travail qui avait démarré le 20 décembre 2018 avec notre regrettée collègue Marielle de Sarnez, qui présidait la commission des affaires étrangères de Nous avions eu l'occasion de vous faire part, monsieur le ministre, d'une série de propositions destinées à alimenter le débat sur la loi d'orientation relative à la solidarité internationale, dont l'examen, à l'époque, nous semblait imminent. Nous voilà donc enfin, deux ans et demi plus tard, arrivés au terme de ce cheminement, certes plus long que prévu, mais nous y sommes parvenus. Et si nous examinons ce projet de loi de programmation relatif au développement solidaire et à la lutte contre force est de constater que ces enjeux sont peut-être encore plus actuels en 2021 qu'en 2018. En effet, l'Afrique a connu en 2020 la pire récession de son histoire, ce qui a plongé des millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Dans tout le continent, la pandémie est aujourd'hui en pleine explosion. Au-delà des initiatives annoncées par la France ou par le G7 pour accélérer l'envoi de vaccins, nous devons redoubler nos efforts en faveur des services de première nécessité : la santé, l'éducation, l'agriculture. Je rappelle que, d'ici à 2050, la population des quatre pays du Sahel va tripler. En 2100, un habitant de la planète sur trois sera africain, tandis que la population de la Chine sera dépassée par celle du Nigéria. Voilà donc le grand défi des prochaines décennies. En outre, le Président de la République a annoncé le 10 juin dernier la fin prochaine- plus exactement, le redéploiement Cela ne signifie pas la fin de tout engagement militaire français dans la région, mais il est clair que notre effort d'aide au développement en faveur du Sahel doit s'intensifier pour devenir désormais notre première arme contre l'extrémisme islamique. Dans ce contexte difficile, le projet de loi que nous devrions adopter définitivement aujourd'hui trace des perspectives très claires. Il nous donne de nouveaux instruments pour aller de l'avant. Le 18 mai dernier, le Sénat adoptait un texte profondément modifié par rapport à celui de l'Assemblée nationale. En commission des affaires étrangères, nous avons clarifié et hiérarchisé les grands objectifs de cette politique afin de la rendre plus compréhensible, plus lisible, pour nos concitoyens. Nourrir, soigner, instruire telles sont les grandes priorités que nous avons souhaité remettre au premier plan afin de mentionner les grands enjeux transversaux que sont la protection de la planète et la défense des droits humains. En concertation avec la commission des finances, et avec son rapporteur pour avis Jean-Claude Requier, que je salue, nous avons également ajouté au texte la programmation financière qui lui faisait cruellement défaut. En outre, nous avons augmenté significativement la part de la taxe sur les transactions financières concourant à cette politique. Soucieux de concentrer les financements sur les pays qui en ont le plus besoin, nous avons inscrit une série de trois cibles relatives aux dons, aux crédits bilatéraux et aux pays prioritaires, en parfaite cohérence avec les grands objectifs que nous avions définis pour cette aide. En commission, puis en séance publique, nous avons également renforcé le rôle du ministre chargé du développement, réaffirmé la tutelle ministérielle sur l'AFD un contrat d'objectifs et de moyens, contrat qui sera rénové et développé avec des dispositions relatives à l'action des ONG. De même, nous avons amélioré la promotion des droits humains dans toutes leurs déclinaisons. Enfin, nous avons introduit un dispositif relatif aux biens mal acquis que nous devons en particulier à la ténacité de notre collègue Jean-Pierre Sueur. Enfin, nous avons modifié la composition de la nouvelle commission d'évaluation, commission qui est un apport essentiel de ce texte. Nous avons souhaité y introduire, c'est vrai, la présence de quatre parlementaires. Un regard pragmatique et soucieux des réalités du terrain, ainsi qu'un lien permanent avec le Parlement, chargé du contrôle des politiques publiques : voilà les raisons qui justifient pleinement notre présence future Nous pouvions d'ailleurs nous prévaloir de l'existence de nombreux organismes de contrôle, d'évaluation ou de régulation dans lesquels la présence des parlementaires a démontré amplement toute sa pertinence et son utilité. Nombre de ces apports du Sénat ont été bien accueillis par les députés : la clarification des objectifs, le ciblage, le renforcement de la gouvernance ou encore les dispositions relatives à la défense des droits humains ont été, pour l'essentiel, confirmés par la Sur la question de la programmation financière et sur celle de la commission d'évaluation, en revanche, ce n'est qu'à l'issue d'une longue et riche discussion que nous avons pu construire les compromis nécessaires.

saluer l'esprit d'ouverture manifesté par mon homologue, Jean-Louis Bourlanges, et par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Hervé Berville, grande conscience, s'il en est, dans ce domaine. Ainsi, sur la question de la programmation financière, nous avons finalement obtenu l'inscription, au sein du texte, d'une trajectoire réaliste pour la période 2023-2025, avec des étapes à 0,61 %, 0,66 % et 0,7 % du RNB consacré à l'aide publique au développement. Le cap est ainsi donné. Il incarne la volonté que nous partageons tous dans les deux assemblées, quelles que soient nos sensibilités, de prendre toute notre part à l'effort de réduction des inégalités mondiales. C'est l'intérêt des populations aidées, mais, nous le savons tous, c'est aussi l'intérêt de la France. S'agissant de la commission d'évaluation, les députés voulaient créer un organisme essentiellement administratif et technique, uniquement composé de professionnels de l'évaluation. Nous restions pour notre part attachés à la présence de parlementaires afin de renforcer le caractère à la fois démocratique et pragmatique de l'évaluation. Alors, nous avons ensemble imaginé- j'ai aidé autant que j'ai pu -une commission composée de deux collèges : le premier constitué d'experts indépendants rendant régulièrement compte et discutant de ses travaux avec le second, qui sera constitué de parlementaires. Au total, le résultat auquel a abouti la commission mixte paritaire nous paraît tout à fait satisfaisant. C'est d'ailleurs aussi parce que, de son côté, le Gouvernement ne s'est jamais montré fermé à la discussion, s'efforçant au contraire de faire progresser le débat. C'est pour cela que nous sommes parvenus à faire émerger ce consensus républicain

de cette législature. Je tiens à vous remercier publiquement pour l'esprit tout à fait convivial, constructif et empreint d'une volonté de dialogue permanent avec lequel vous avez conduit ce projet. J'y vois votre

La France, mes chers collègues, n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est généreuse. Avec une dimension peut-être plus forte encore, nous avons aujourd'hui le sentiment d'agir pour la paix. La discussion générale est la commission mixte paritaire. Je rappelle que,en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Deuxièmement, la mention du représentant des pays partenaires fait allusion à une phrase qui n'existe plus dans la version finale de l'article 9. En revanche, un tel membre pourra bien entendu être nommé parmi les dix membres auxquels il est fait référence plus haut dans l'article. Quel est l'avis du

Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, juste un mot après ce vote à l'unanimité du Sénat, qui fait suite à un même vote unanime de l'Assemblée nationale. J'en conçois une certaine fierté pour la France ce vote, vos votes font honneur à notre pays, à ses valeurs, à la place qu'il occupe dans le monde. Je parlais tout à l'heure d'une certaine idée française de la solidarité : vous en avez marqué une étape supplémentaire et donné beaucoup de force à notre action dans le monde. Je voulais vous en remercier et vous redire ma fierté.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est parvenue hier à un texte commun sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Cet accord, qui est le fruit d'échanges nourris avec nos collègues députées Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean, auteures du texte et rapporteures pour l'Assemblée nationale, répond globalement aux attentes et aux préoccupations exprimées par le Sénat. Il devrait nous conduire à adopter, une dernière fois en ce qui nous concerne, cette proposition de loi. Le renforcement de la démarche d'évaluation et de prévention des risques professionnels au sein des entreprises est un objectif que nous partageons tous. Nous avons cependant tenu à l'aborder avec pragmatisme, en garantissant notamment le caractère opérationnel de l'élaboration et de la conservation et de la conservation du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). Je me félicite en particulier que l'obligation de dépôt dématérialisé du DUERP, introduite par le Sénat à l'article 2, soit maintenue dans le texte de la Sa mise en oeuvre sera bien entendu échelonnée dans le temps pour tenir compte de la taille des entreprises et de leurs contraintes, et nous confions le soin aux organisations patronales de définir les modalités du déploiement du portail numérique qui centralisera ce dépôt dématérialisé. Nous partagions par ailleurs avec les rapporteures de l'Assemblée nationale le souci d'améliorer la qualité des prestations des services de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) et leur mobilisation dans l'ensemble de leurs missions, dans une logique de service rendu aux entreprises adhérentes et à leurs salariés. À l'article 8, qui contient plusieurs avancées concernant le cadre d'exercice des SPSTI, la rédaction finale reprend plusieurs apports du Sénat : la précision apportée à la définition de l'ensemble socle de services l'initiative donnée aux partenaires sociaux, à travers une proposition du comité national de prévention et de santé au travail (CNPST), pour élaborer le cahier des charges de la nouvelle procédure de certification enfin, l'introduction d'un régime d'administration provisoire permettant de remédier à une situation de dysfonctionnement grave d'un SPSTI qui l'empêcherait d'assurer ses missions. Nous avons également défendu l'application à l'ensemble des SPSTI, à l'article 13, d'une obligation de mise en conformité de leurs systèmes d'information et de leurs outils numériques à des référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Concernant la tarification de ces services, le Sénat a introduit à l'article 9 deux modifications importantes : d'une part, l'encadrement du montant des cotisations dans un « tunnel » défini par référence au coût moyen national de l'offre socle d'autre part, le calcul des cotisations en fonction du nombre de personnes suivies non proratisé en équivalent temps plein (ETP). Ces dispositions, qui traduisent les ambitions de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre dernier en matière de transparence financière des SPSTI et permettent d'assurer une meilleure équité entre les entreprises, sont reprises dans leur rédaction issue du Sénat. En matière de suivi et d'accompagnement des travailleurs vulnérables, le Sénat avait veillé à poursuivre avec un souci d'efficacité et d'opérationnalité l'objectif d'améliorer les outils de maintien dans l'emploi des personnes malades ou handicapées. mixte paritaire reprend certaines des améliorations apportées par le Sénat au dispositif de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui doit être créée dans chaque SPSTI la possibilité de mutualiser la cellule, ainsi que la fixation dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'exigences minimales sur sa composition. S'agissant, à l'article 18, du rendez-vous de liaison qui peut être organisé entre un travailleur en arrêt de travail de longue durée et son employeur, nous avons abouti à une rédaction intermédiaire qui rétablit la participation du SPSTI à ce rendez-vous, ainsi que l'avait prévu l'Assemblée nationale, mais maintient la possibilité, introduite par le Sénat, que l'employeur le sollicite. En matière de suivi de certains publics particuliers, plusieurs apports du Sénat figurent dans le texte de la l'expérimentation d'actions de prévention collective destinées aux salariés intérimaires, à l'article 17 A ; les modalités de mise en oeuvre du suivi de l'état de santé des salariés du particulier employeur, à l'article 17 la possibilité donnée au chef d'entreprise de bénéficier des services du SPSTI auquel son entreprise est affiliée, à l'article 17.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je me réjouis à mon tour que la commission mixte paritaire soit parvenue à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Cet accord conclut des échanges fructueux entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour l'élaboration du texte qui vous est soumis aujourd'hui. Il concrétise une démarche inédite de démocratie sociale et parlementaire au service de la protection de la santé des travailleurs. Il me semble que la commission mixte paritaire est parvenue à un texte équilibré qui retient d'importants apports du Sénat. Nous avons veillé à réunir les conditions d'une médecine du travail moderne, au service de la prévention et adaptée aux nouveaux défis posés par l'évolution des technologies et des modes d'organisation du travail. Nous nous sommes accordés, avec nos collègues députés, sur le fait que l'évaluation des risques professionnels ne devait pas être perçue comme une contrainte administrative subie par les entreprises. Au contraire, les employeurs doivent saisir l'occasion de cette évaluation, qui engage leur responsabilité, pour répondre à leur obligation de sécurité à l'égard de leurs salariés. Pour sa diffusion effective dans l'ensemble des entreprises et sa déclinaison en actions de prévention concrètes, cette évaluation doit être adaptée à la réalité du fonctionnement des entreprises. C'est pourquoi le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire reprend, à l'article 2, les apports du Sénat visant à adapter les modalités de définition du plan d'actions de prévention, afin que celles-ci soient proportionnées aux enjeux et aux moyens internes des entreprises, notamment les TPE et PME de moins de cinquante salariés. Avec ma collègue rapporteur Pascale Gruny, nous avons plaidé pour le décloisonnement de la médecine du travail et de la santé publique, nécessité que nous avions identifiée dès la rédaction de notre rapport d'information sur la santé au travail d'octobre 2019. C'est pourquoi le renforcement, à l'article 2 , du suivi post-exposition des travailleurs exposés à des risques particuliers, ainsi que l'approfondissement de la coopération entre la médecine du travail et la médecine de ville constituent, à mon sens, des avancées significatives qui ont été approuvées par la Cette coopération renforcée doit se traduire par un meilleur partage d'informations entre professionnels de santé dans un objectif de prévention et de coordination des parcours, que ce soit au travers du dossier médical partagé, du dossier médical en santé au travail ou du recours aux consultations à distance. Décloisonnement ne veut pas dire pour autant uniformisation : par sa connaissance fine des entreprises, la médecine du travail reste la mieux placée pour assurer le suivi médical des travailleurs. Nous avons ainsi défendu avec ma collègue Pascale Gruny la spécificité de la médecine du travail, dont l'attractivité doit être considérablement renforcée. L'expérimentation introduite par le Sénat à l'article 21 permettant d'étendre dans trois régions le droit de prescription des médecins du travail des médecins du travail constitue un premier pas en ce sens. De nombreux efforts restent à mener pour attirer davantage les étudiants en médecine vers cette spécialité. J'invite à cet égard le Gouvernement à revoir les conditions de stage des externes de médecine pour leur permettre de se familiariser aux enjeux de la médecine du travail. Ils auraient alors une meilleure appréhension de ces sujets lors de leur choix de spécialité pour l'internat. Un médecin généraliste ne pourra pas remplacer un médecin du travail, d'autant que les difficultés de démographie médicale touchent particulièrement ces deux spécialités. Dans ce contexte, nous considérons que le dispositif de médecin praticien correspondant constitue un moyen de susciter des vocations chez des médecins généralistes qui seraient tentés, par exemple en milieu de carrière, par un exercice salarié en médecine du travail, même s'il ne résoudra pas à lui seul les tensions démographiques que connaissent les services de santé au travail. En outre, la montée en compétences cliniques des infirmiers de santé au travail est une piste prometteuse. Ces professionnels vont prendre une place croissante dans le suivi de la santé des travailleurs et la qualité de leur formation devra être garantie. Enfin, sur la question plus périphérique, mais non moins importante, de la définition du harcèlement sexuel au travail, à l'article 1, le texte de la commission mixte paritaire conserve, moyennant un ajustement purement rédactionnel, la modification apportée par le Sénat sur l'initiative de nos collègues Laurence Cohen et Laurence Rossignol, qui vise à centrer cette définition sur les faits subis par la victime et non sur l'intention de l'agresseur. C'est donc un texte équilibré, répondant à l'objectif d'une meilleure prévention en santé au travail de l'ensemble des travailleurs et intégrant des apports significatifs du Sénat que nous vous proposons d'adopter. La parole est à M.

je suis heureux de prendre la parole devant vous à l'occasion de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail.

Votre travail de grande qualité permet d'aboutir aujourd'hui à un texte solide et équilibré qui, conformément à l'engagement du Gouvernement, vient donner une réalité législative et démocratique à l'accord national interprofessionnel conclu entre les partenaires sociaux en décembre dernier. Je me félicite de cette complémentarité liant à la vitalité de notre dialogue social celle de notre démocratie représentative, dans l'intérêt et pour le bénéfice de la santé de millions de salariés et de leurs employeurs. La crise sanitaire que nous continuons de traverser nous rappelle chaque jour l'enjeu essentiel qu'est l'amélioration de la santé au travail, enjeu pour lequel le Gouvernement est pleinement mobilisé. C'est également une attente forte des salariés et des entreprises que j'ai pu mesurer à travers mes nombreux déplacements depuis plus d'un an à leurs côtés et au sein des services de santé au travail. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous le disais, cette proposition de loi contient de très belles avancées que le Gouvernement soutient. Je ne reviendrai pas dans le détail sur chacune des dispositions, mais j'en résumerai brièvement l'esprit et la teneur.

des obligations proportionnées à leur taille et à leurs moyens, notamment en ce qui concerne les entreprises de moins de cinquante salariés. Le dépôt des documents uniques et leur conservation sur un portail numérique géré par les organisations professionnelles est aussi une avancée importante

De même, le Gouvernement se félicite de l'accord trouvé entre les deux assemblées sur l'accès au dossier médical partagé (DMP) et au dossier médical en santé au travail Je salue également les ajustements apportés sur le rendez-vous de liaison qui permettront de renforcer l'efficacité de ce dispositif destiné à anticiper et à préparer la reprise d'activité du salarié, ainsi que la définition d'un cadre pour la santé au travail des salariés des particuliers employeurs et des assistants maternels, qui permettra de mettre en place, dans le cadre d'un dialogue social de branche, la prise en charge effective de ces publics.

sur le sujet a été rappelé. Pour conclure, comme j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler, le retour d'expérience de la crise du covid-19 doit nous permettre de construire ensemble un modèle de santé au travail plus proche de l'entreprise et des salariés et plus orienté vers l'accompagnement et le conseil pour la mise en place de mesures de prévention collective. Il est en effet essentiel de moderniser notre système de santé au travail afin de l'adapter et de répondre aux enjeux des parcours professionnels du XXI siècle. Le Gouvernement et l'ensemble Le Gouvernement et l'ensemble des acteurs y sont prêts. C'est pour cette raison, et dans l'esprit de consensus qui nous a animés tout au long du débat parlementaire, que je vous invite à suivre les conclusions de la commission mixte paritaire et à voter la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail qui vous est soumise aujourd'hui.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

fruit d'un long processus de démocratie sociale et parlementaire. Mes chers collègues, notre mission était de veiller à ce que la transcription dans la loi de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 9 décembre dernier respecte aussi bien son contenu que son équilibre. Aussi, je me réjouis que la commission mixte paritaire ait trouvé hier un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail, initiée par les députées LaREM, Mmes Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole Grandjean.

apportées, notamment l'adaptation, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, des actions de prévention et de protection découlant du document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels. En gardant la possibilité de réaliser une consultation à distance, sans pour autant utiliser le terme inadéquat de « téléconsultation » ou encore en donnant la possibilité au médecin du travail de ne pas être l'unique animateur et coordinateur de la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle, a tenu compte des modifications que nous avions apportées au texte en séance. La rédaction définitive retient également l'expérimentation d'actions de prévention collective destinées aux salariés intérimaires et la possibilité, pour un chef d'entreprise, de bénéficier du suivi médical assuré par le service de prévention et de santé au travail. Enfin, nous sommes satisfaits que plusieurs des modifications que nous avions défendues en séance aient été conservées, la possibilité de mutualisation des services de santé au travail pour les travailleurs ayant une pluralité d'employeurs, à l'article 17 , ou encore les précisions apportées concernant les infirmières de santé au travail exerçant leurs missions au sein du service de santé des gens de mer, à l'article 23. Une fois de plus, nous pouvons nous féliciter du fonctionnement d'un bicamérisme équilibré, dans lequel chaque chambre a pu faire valoir son point de vue afin d'enrichir le texte de manière constructive.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la commission mixte paritaire sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail a réussi à se mettre d'accord hier après-midi sur un texte au rabais- il Alors que les organisations syndicales et les associations plaidaient en faveur d'une loi qui fasse de la prévention des risques professionnels une priorité, qui garantisse un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail et qui favorise le maintien dans l'emploi des salariés vulnérables, le compte n'y est pas. Bien au contraire, le texte renvoie la responsabilité de la santé et de la sécurité sur chaque salarié, avec la création du passeport de prévention. La proposition de loi remet en cause la visite de préreprise, en court-circuitant le médecin du travail avec les fameux « rendez-vous de liaison Le Gouvernement tente d'effacer le lien de subordination entre les salariés et l'employeur. Seuls les médecins du travail ont la formation et l'indépendance nécessaires pour connaître des raisons personnelles et médicales qui conduisent les salariés à arrêter de travailler. Alors que l'accès à la médecine du travail demeure toujours aussi compliqué sur les territoires, le Gouvernement préfère créer des médecins praticiens correspondants et déléguer des fonctions aux infirmiers, plutôt que de revaloriser les métiers et d'augmenter les salaires. L'expérimentation du droit de prescription des médecins du travail est une revendication des praticiens. C'est une avancée, mais elle n'est pas suffisante pour créer une dynamique sur une filière délaissée depuis des années. La commission mixte paritaire a conservé la proposition du Sénat de créer un portail numérique pour archiver le document unique d'évaluation des risques. Nous étions intervenus contre cet archivage géré par les seules organisations patronales, sans aucune garantie de sécurité pour les données de santé numérisées. La traçabilité des expositions aux risques professionnels doit relever d'un organisme public indépendant, comme les caisses La seule modification positive concerne l'adoption de l'amendement du groupe CRCE présenté par ma collègue Laurence Cohen, qui visait à revenir sur la définition du harcèlement. Les organisations féministes nous avaient interpellés pour maintenir une définition du harcèlement qui permette aux victimes d'obtenir réparation aux prud'hommes, indépendamment de la procédure devant la juridiction pénale. Concernant la majorité des problématiques de santé au travail, les questions demeurent sans réponse. Les salariés devront donc encore patienter avant de bénéficier d'une politique de prévention primaire des risques professionnels qui prenne en compte la pénibilité des postes et l'usure professionnelle. Les millions de salariés en télétravail

Les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste voteront contre cette proposition de loi. La parole

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail n'est pas un texte à destination exclusive des professionnels des ressources humaines. Il nous concerne tous, c'est un texte de société. La santé au travail, dans sa dimension de réparation comme de prévention, est un enjeu essentiel ; confrontée à des défis majeurs, elle ne doit pas rester sous les radars. La pénurie de professionnels de santé, la crise sanitaire inédite, le développement d'autres méthodes de travail, comme le télétravail, les reconversions professionnelles, mais aussi la très grande hétérogénéité du monde de l'entreprise et de l'offre des services de santé au travail ont amené les partenaires sociaux à travailler conjointement sur ces sujets. Ils ont conclu, le 9 décembre dernier, un accord national interprofessionnel qui s'appuie sur de récents travaux parlementaires, en particulier ceux de nos collègues Pascale Gruny et Stéphane Artano. Le texte Le texte législatif qui en a découlé a été adopté par l'Assemblée nationale le 17 février dernier, puis modifié par le Sénat le 6 juillet. La difficulté, pour la commission mixte paritaire qui s'est réunie hier, ne fut pas de trouver un consensus sur les trente-huit articles restant en discussion. La volonté conjointe d'aboutir était là, les sujets maîtrisés et approfondis, les apports des deux chambres furent pris en compte dans une synthèse heureusement conclusive. Non, la difficulté, à mon sens, fut pour nous de garder constamment comme objectif de produire un texte utile, opérationnel, adapté, que la culture de la prévention du risque puisse ainsi se diffuser, y compris au sein des très petites entreprises, sans être vécue comme punitive, alors que se profile dans certains secteurs une pénurie de main-d'oeuvre.

permettent aux entreprises de moins de cinquante salariés de définir une liste d'actions de prévention des risques et de protection dans leur document unique d'évaluation des risques professionnels, sans formalisme supplémentaire

organisent l'accès réciproque et circonscrit à des données contenues dans le dossier médical partagé et dans le dossier médical en santé au travail, en veillant toujours au strict respect du secret médical et au recueil du consentement libre et éclairé du salarié. du travail la possibilité de déléguer l'animation et la coordination de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle à un membre de l'équipe pluridisciplinaire qui agit sous sa responsabilité

également une visite médicale de mi-carrière et précise les complémentarités entre suivis de santé en ville et au travail. Ces deux spécialités médicales connaissant la même situation de pénurie, le médecin d'aptitude reste bien le médecin du travail, un spécialiste irremplaçable. confirme qu'une formation spécifique doit être dispensée avant 2023 aux futurs infirmiers de santé au travail, qui occupent un rôle de plus en plus central au sein des services de santé au travail. enfin, aux médecins du travail la possibilité de déléguer l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire, laquelle reste toutefois toujours sous leur responsabilité. Mes chers collègues, en conclusion de ces travaux, je souhaite également souligner l'intérêt qui a été porté, au-delà des salariés, aux chefs d'entreprise

la montée en puissance de la prévention en santé au travail partout et pour tous, sans alourdir la charge de travail de ces professionnels de santé, de plus en plus rares. Nous avons refusé d'acter le déclin d'une spécialité médicale à part entière, préférant placer nos espoirs dans des mesures qui la rendraient plus attractive.

Que chacun, employeur et salarié, trouve là des pistes de progrès gagnant-gagnant, des outils pratiques qui permettent de protéger ce bien unique et irremplaçable qu'est la santé de nos collaborateurs. Vous l'aurez compris, les centristes voteront ce texte. La parole est

en proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail. Nous regrettons que les médecins du travail n'aient pas été plus largement associés à la concertation avec les partenaires sociaux. Ils sont pourtant bien placés pour évaluer la santé au travail et pour agir en faveur de son amélioration et de la prévention. Faute d'un accord ambitieux et de ce cadre contraint, accentué par l'application stricte des articles 40 et 45 de la Constitution, nous n'obtenons au final qu'une proposition de loi.

Les versions issues de l'Assemblée nationale et du Sénat étaient insatisfaisantes et nous ne constatons pas d'amélioration significative du texte dans la rédaction de la commission mixte paritaire. présente au contraire un risque de dégradation de la protection des salariés. Le texte opère un véritable glissement de la santé au travail vers des missions de santé publique et de promotion de la santé globale, soit une dilution de la mission de santé au travail au profit de la notion de santé en entreprise. Il y a une véritable confusion entre la santé au travail, c'est-à-dire la santé relative à l'organisation du travail en matière de prévention des risques primaires, et la santé individuelle des travailleurs, relative aux comportements vis-à-vis par exemple de l'alcool, du tabac ou de la pratique sportive. commission mixte paritaire supprime la disposition introduite par le Sénat précisant que le personnel de santé au travail contribue à la sensibilisation aux violences conjugales ou sexuelles. Le rapprochement entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, voulu dans ce texte, ne s'applique pas dans le cas des violences intrafamiliales, pourtant grande cause du quinquennat. Nous regrettons très fortement que ce sujet soit passé à la trappe de la Cette proposition de loi présente un risque pour les travailleurs, en organisant la déresponsabilisation de l'employeur en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés. L'instauration d'un passeport de prévention à l'article 3 peut être perçue, en réalité, comme un permis autorisant les employeurs à se dégager de leurs responsabilités en matière de sécurité, au motif qu'un travailleur a été préalablement informé et formé. mixte paritaire n'a malheureusement pas apporté de solution à ce problème, pointé par notre groupe lors des débats au Sénat. Par ailleurs, donner accès au dossier médical partagé au médecin du travail représente un danger pour la protection des salariés. Cet accès au dossier médical peut leur être préjudiciable, en particulier lors des visites d'embauche et de reprise du travail, surtout lorsqu'il y a une nécessité d'adaptation à l'emploi.

Toutefois, les discussions entre les députés, les sénateurs et le Gouvernement ont permis quelques évolutions positives du texte. La première est la prise en compte aussi bien des agissements sexistes que des propos ou comportements à connotation sexuelle dans les situations visées dans la définition du harcèlement sexuel au travail. La prise en compte des faits subis par la victime, indépendamment de l'intention des personnes concernées de les imposer, va dans le sens des propositions que nous avions formulées lors de l'examen au Sénat. Par ailleurs, nous saluons l'adoption d'un amendement à l'article 2 visant à instaurer un suivi renforcé pour les salariés ayant été exposés à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. De même, la nouvelle version du texte consacre une vigilance spécifique quant aux nouvelles formes d'organisation du travail, en particulier au télétravail. Elle dispose que les services de prévention et de santé au travail prêtent une attention particulière à l'impact que peut avoir le télétravail sur la santé et la sécurité des travailleurs. Dans le même sens, nous sommes également favorables au rétablissement de la disposition retenue par l'Assemblée nationale selon laquelle le service de prévention et de santé au travail devra être associé au futur rendez-vous de liaison entre l'employeur et le salarié en arrêt de travail. Cette présence permet de protéger le salarié des éventuelles pressions de l'employeur et d'éviter un tête-à-tête entre eux. S'agissant de la possibilité pour les infirmiers disposant de la qualification nécessaire d'exercer en pratique avancée en matière de prévention et de santé au travail, la disposition ne nous satisfait pas totalement. Si elle permet, en effet, de protéger les infirmiers, qui exercent sous la responsabilité du médecin du travail, elle empêche toutefois le plein exercice de la pratique avancée et risque de dévaloriser le métier d'infirmier et cette spécialisation. Cette proposition de loi, porteuse de grands espoirs concernant la pénurie de médecins du travail, la prévention des risques primaires et la lutte contre les inégalités territoriales, n'apporte en réalité pas de réponse concrète aux difficultés posées par l'exercice de la médecine du travail.

a repris un certain nombre des avancées apportées par le Sénat en première lecture. Je félicite Mme et M. les rapporteurs pour leur travail qui a permis d'améliorer le texte. Je soutiens les mesures adoptées visant à adapter les actions de prévention aux entreprises de moins de cinquante salariés, ainsi que le dépôt du document unique d'évaluation et de prévention des risques professionnels sur un portail numérique pour garantir sa conservation. Je suis favorable à la valorisation du rôle du médecin du travail à travers l'expérimentation d'une extension de son pouvoir de prescription dans les limites des missions de prévention. Dans le cadre de la crise sanitaire, les médecins du travail ont déjà la possibilité de prescrire des arrêts de travail. Le texte étend cette possibilité à la prescription des soins ou des examens nécessaires à la prévention de l'altération de l'état de santé des salariés. par la commission mixte paritaire : les salariés intérimaires pourront bénéficier d'actions de prévention collective. Près de trois millions de salariés verront ainsi leur accès à la santé renforcé. Le texte conforte, par ailleurs, le suivi de l'état de santé des salariés des particuliers employeurs et des chefs d'entreprise, qui pourront bénéficier du suivi assuré par le service de prévention et de santé au travail auquel adhère leur entreprise. Les récentes enquêtes réalisées auprès de dirigeants de TPE et de PME témoignent d'une forte détérioration de leur état de santé en raison de la crise sanitaire, avec des risques particulièrement élevés de burn-out. La proposition de loi améliore la coordination entre médecine du travail et médecine de ville et favorise la délégation de compétences aux infirmiers en pratique avancée, sous la responsabilité du médecin. praticiens correspondants, qui pourront se former en médecine du travail, contribuera à renforcer les effectifs de médecins du travail dans les territoires sous-dotés,

essentiel d'organiser une plus grande fluidité des parcours entre médecine de ville et médecine du travail et de valoriser cette profession. Ce texte propose des avancées, la commission des affaires sociales du Sénat y a largement contribué et notre groupe se félicite du travail collégial mené avec l'Assemblée nationale dans le cadre de la

santé au travail ambitieux, plutôt qu'une transcription incomplète de l'accord national interprofessionnel de 2020, qui n'en respecte même pas tous les équilibres, au détriment des salariés. Non seulement le texte n'est pas à la hauteur des enjeux, mais il poursuit la démédicalisation de la santé au travail. Il ne revient pas sur la dégradation des services de santé au travail issue des réformes antérieures, et, par certains de ses dispositifs, l'aggrave, comme il n'écarte pas le risque d'échappement de la responsabilité personnelle de l'employeur quant à ses obligations en termes de santé et de sécurité. Pendant les débats, les écologistes ont porté une autre vision du travail et de la santé au travail. En intimant au Parlement de se contraindre au respect de l'accord interprofessionnel signé par quatre syndicats, la majorité présidentielle a dénié à l'État et au Parlement leur responsabilité propre quant à la santé au travail. Beaucoup de nos propositions ont été rejetées, rejetées, y compris celles qui avaient été coconstruites avec les professionnels et les syndicats, dont certains avaient pourtant signé l'ANI. Le résultat est encore aggravé au sortir de la commission mixte paritaire.

car, si le pouvoir d'organisation n'est pas partagé, alors la responsabilité ne saurait l'être ; or le texte consacre des dispositifs qui la relativisent. Nous voulions mettre en lumière les risques psychosociaux, deuxième cause d'arrêts de travail

le texte confirme l'accès au dossier médical partagé pour les professionnels des SPST et balaye le renforcement du consentement du salarié, pourtant adopté en commission au Sénat. Nous avions combattu les dispositifs qui actent l'effacement des médecins du travail et déprécient leur spécialité. Ainsi, le texte prévoit le recours à des médecins de ville correspondants pour le suivi des salariés. Nous souhaitons

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d'un an nous rappelle combien la santé au travail a légitimement sa place au sein de notre politique de santé publique. nombreuses sont les études mettant en évidence les limites de l'organisation des services médicaux du travail. Je pense notamment au rapport d'information publié il y a deux ans déjà par nos deux rapporteurs, Pascale Gruny et Stéphane Artano, que je tiens Les deux dernières grandes réformes de la santé au travail, menées en 2011 et en 2016, ont certes apporté certaines améliorations, mais force est de reconnaître qu'il est aujourd'hui nécessaire de faire davantage reposer la santé au travail sur une logique de prévention et non plus seulement sur des mécanismes de réparation des atteintes à la santé des travailleurs.

preuve que nos deux assemblées savent s'entendre sur un sujet essentiel pour la vie de nos concitoyens et de nos travailleurs. Pour ma part, je regrette

Beaucoup a déjà été dit par les orateurs précédents ; je ne reviendrai donc que brièvement sur les points de ce texte qui constituent des avancées, comme l'expérimentation du droit de prescription des médecins du travail, chère à notre collègue rapporteur Stéphane Artano. Selon ses propres termes, elle constitue une réponse au défi de la démographie médicale, mais elle nous offre aussi l'occasion de décloisonner médecine de ville et médecine du travail, dans un même effort de cohérence en santé publique.

conservé l'obligation de dépôt dématérialisé du DUERP sur un portail numérique géré par les organisations d'employeurs, ainsi que l'expérimentation d'actions de prévention collective destinées aux salariés intérimaires.

Considérant que ce texte représente une avancée, même s'il n'est pas parfait, et qu'il donne à la médecine du travail les moyens de s'ouvrir à une approche pluridisciplinaire

La proposition de loi que nous nous apprêtons à adopter est en effet le fruit de riches mois d'un travail d'abord syndical, puis parlementaire. Pour répondre aux défis actuels en matière de santé au travail, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord national interprofessionnel le 9 décembre dernier. Ensuite, dans un format peu commun, le Parlement a été saisi de ce texte d'origine syndicale. L'exercice n'est pas toujours simple : sans rien renier de notre pouvoir souverain de voter la loi, il nous a fallu trouver un équilibre qui respecte la volonté des organisations professionnelles. Je crois que nous y sommes arrivés ; je tiens à saluer à cette tribune, avec force, le travail de fond accompli par nos deux rapporteurs, Pascale Gruny et Stéphane Artano. Le texte qui sera bientôt gravé dans le marbre de notre droit apporte des réponses circonstanciées à des problèmes que la crise sanitaire a contribué à mettre en lumière. En renforçant la prévention dans le milieu professionnel, les entreprises seront demain plus à même de détecter en amont des pathologies qui nécessitent une prise en charge rapide. Il convenait pour cela de muscler certains dispositifs, d'en rationaliser d'autres, voire d'en créer de nouveaux. C'est ainsi que le document unique d'évaluation des risques professionnels deviendra bientôt la pierre angulaire de cette prévention, la référence stratégique permettant de recenser les risques internes à l'entreprise et les actions que celle-ci doit mettre en oeuvre pour les pallier. à ce texte, médecine du travail et médecine de ville seront un peu moins cloisonnées et un peu plus complémentaires, grâce notamment à l'ouverture facilitée de l'accès au dossier médical partagé et au dossier médical en santé au travail.

Des critiques visaient l'hétérogénéité de ces offres de manière récurrente ; je crois que la procédure de certification que nous allons adopter permettra d'y mettre bon ordre, de même que la distinction entre offre socle et offre complémentaire. Enfin, cette proposition de loi va permettre à de nouveaux publics, comme les personnes en situation de handicap, de bénéficier d'une couverture préventive complète, ce qui n'est au fond qu'une mesure de bon sens. Mes chers collègues, le dialogue parlementaire a porté ses fruits ; je me réjouis du maintien dans le texte élaboré par la commission mixte paritaire de nombreuses dispositions introduites sur l'initiative de notre assemblée. C'est le cas tout d'abord de l'équilibre trouvé entre la nécessaire exigence de prévention de la santé au travail et la volonté de ne pas alourdir les contraintes pesant sur les très petites entreprises. Notre commission des affaires sociales a ainsi prévu que les entreprises de moins de cinquante salariés pourraient définir leurs actions de prévention sans se voir imposer le formalisme d'un programme annuel de prévention. C'est une rédaction de compromis qui a été retenue elle vise à garantir que les actions de prévention et de protection que les entreprises de moins de cinquante salariés doivent définir seront obligatoirement listées dans le DUERP. a, par ailleurs, maintenu l'ouverture de l'offre socle de services fournis par les SPST aux travailleurs indépendants, que le Sénat avait introduite en première lecture. Notre assemblée a enrichi sur de nombreux autres points encore le texte de l'ANI examiné préalablement à l'Assemblée nationale. Nous avons ainsi souhaité renforcer l'approche préventive de la santé au travail, grâce à la prise en compte des situations de polyexpositions pour les travailleurs exposés à des risques chimiques, définir plus précisément l'offre socle de services délivrés par les SPST, enrichir les dispositions concernant la certification et la tarification des mesures mises en place par les services de prévention ou encore mieux inclure les questions de harcèlement sexuel dans les politiques de prévention. Je pourrais également citer le compromis trouvé avec nos collègues députés concernant l'intégration du passeport de prévention au passeport de formation, lorsque les salariés disposent d'un tel document, mais aussi l'amélioration du dispositif de visite de mi-carrière

Mes chers collègues, comme vous le constatez, beaucoup de mesures adoptées par notre assemblée figurent dans le texte final ; c'est une réalité dont nous pouvons nous réjouir. Dans l'intérêt des salariés et des entreprises, je souhaite donc que les dispositions réglementaires puissent être prises rapidement afin d'assurer une couverture préventive optimale à tous les employés de notre pays.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, mesdames les rapporteures, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, depuis le début, le projet de loi que vous examinez est un texte que nous avons voulu équilibré et profondément républicain. C'est en tout cas un texte nécessaire, d'une grande évidence et, en même temps, d'une ambition forte et inédite. Une grande évidence, parce que ce texte encadre et accompagne mieux le monde associatif, en interdisant le financement public de structures ou d'organismes qui rejettent nos valeurs et parce qu'il donne à l'État, sous le contrôle étroit du juge des libertés, des moyens plus efficaces pour mettre un terme aux activités associatives qui menacent gravement la paix publique. agit concrètement pour la dignité humaine, en mettant au ban des pratiques qu'il ne devrait même plus être nécessaire d'exclure tant elles heurtent ce qui constitue notre vision commune de la dignité de la personne humaine. Ce texte renforce notre arsenal dans le combat sans relâche que nous voulons mener contre les discours et les agissements de haine. Ce texte nous donne un droit de regard sur les structures et les salariés qui enseignent à nos enfants, afin de s'assurer que l'éducation ne servira jamais de cheval de Troie à un projet séparatiste, de quelque obédience qu'il provienne. rappelle utilement la liberté si essentielle qu'est la liberté de culte, qui doit toujours s'exercer dans la légalité républicaine et s'inscrire dans un cadre, où garanties et avantages s'équilibrent harmonieusement. Enfin, ce texte affirme sans hésitation que la neutralité et la laïcité doivent s'appliquer aux délégataires de service public.

Nous affirmons avec force qu'il n'est pas possible de menacer des fonctionnaires pour que le service public se plie à des exigences communautaristes ou séparatistes. Nous réaffirmons avec force la portée des principes de neutralité et de laïcité, y compris dans les collectivités locales avec le référent laïcité. Nous avançons dans la protection des personnes contre la haine sans visage que l'on peut trop souvent trouver sur internet, notamment sur les plateformes et les réseaux sociaux. fait, personne n'avait encore affirmé avec autant de clarté la nécessité du respect par tous et toutes des règles de la République. Enfin, nul texte n'avait osé faire évoluer la loi de 1905, tout en restant fidèle à l'esprit et à la volonté de ses rédacteurs. Nul texte n'était parvenu à exprimer à la fois le caractère unique du culte et la nécessaire adaptation de ce cadre à la réalité de notre société française du XXI siècle.

Ce texte a été longuement examiné par votre Haute Assemblée. Les débats parlementaires ont permis de l'enrichir, parfois de le renforcer. Aussi, nous avons retenu et valorisé des apports sénatoriaux qui allaient dans le sens de l'équilibre souhaité par le Gouvernement. Compte

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui en nouvelle lecture un texte dont chacun s'accorde à penser qu'il est regrettable qu'il n'ait pas fait l'objet d'un accord entre les deux chambres. Pourtant, sans surprise, le refus de tout compromis de l'Assemblée nationale, qui avait conduit à l'échec de la commission mixte paritaire, n'a fait que se confirmer à l'issue de la nouvelle lecture par les députés. À l'issue des travaux du Sénat, 129 articles restaient en discussion. L'Assemblée nationale en a adopté 23 sans modification ; elle a supprimé 39 des 56 articles ajoutés par notre assemblée.

Elle n'a retenu aucun des dispositifs d'encadrement présentés par notre commission de la culture pour éviter les dérives séparatistes, tout en préservant la liberté d'enseignement. Elle n'a pas plus retenu les dispositions tendant au respect du principe de neutralité dans l'enseignement supérieur ni l'essentiel des dispositions adoptées par le Sénat sur le sport- c'est un vrai regret. S'agissant des travaux de notre commission des lois, l'Assemblée nationale a supprimé l'obligation de neutralité pour les accompagnateurs scolaires, l'interdiction des listes communautaires ou encore l'interdiction de faire figurer

Notre souhait de marquer clairement le cadre de notre vivre ensemble et la nécessité d'exclure les pressions religieuses n'a donc pas été entendu. Il en a été de même pour la police des cultes, où l'Assemblée nationale a largement rétabli son texte, tout en retenant notre volonté de maintenir la responsabilité accrue du ministre des cultes et l'article qui la fonde au sein de la loi de 1905. À l'inverse, malgré les doutes sérieux que nous avons exprimés sur l'efficacité des mesures proposées, nationale a rétabli des dispositions présentées comme devant protéger les femmes. Certes, quelques avancées du Sénat ont été retenues ; je pense notamment à l'obligation d'obtenir un avis du préfet sur les projets relatifs à des constructions destinées à l'exercice du culte, adoptée sur l'initiative de notre collègue Philippe Dallier, et à certains amendements de nos collègues Roger Karoutchi, Valérie Boyer, Jean-Pierre Grand ou Jean Sol. Néanmoins, ces apports sont faibles au regard de nos divergences. Pourtant, lorsque le Président de la République, le 28 mars 2018, dans la cour des Invalides, devant le cercueil d'Arnaud Beltrame, appelait à combattre l'hydre islamiste, les Français ont cru entendre une vraie volonté politique de lutter contre le séparatisme.

Or force est de constater que trois ans plus tard, en ce mois de juillet 2021, le texte tant attendu n'apportera- hélas ! -aucune réponse politique à ce qui menace notre pays : l'entrisme islamiste. mots, si je puis dire, mais pas d'actes, ni même probablement de volonté affirmée de lutter. Quand une loi censée préserver le respect des principes de la République ne fixe pas clairement la manière avec laquelle elle imposera un cadre et des règles à celles et ceux qui veulent faire valoir leur idéologie religieuse et fragiliser la République une, indivisible et laïque, l'inquiétude légitime de la plupart des citoyens de ce pays ne risque pas d'être apaisée.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, tout en partageant les objectifs du texte, le Sénat a cherché à trouver un équilibre entre la défense des principes de la République et la liberté religieuse, qui s'exerce notamment par le libre exercice du culte et par la possibilité de créer des associations cultuelles. Il ne fait aucun doute que la loi doit être la même pour tous et que l'on ne peut distinguer entre les cultes qui seraient intégrés à la République et ceux qui devraient encore faire la preuve de leur intégration. La volonté de faire prévaloir une idéologie sur les lois de la République au nom de la religion n'est pas propre à un seul courant spirituel, mais la protection des libertés implique que les contraintes administratives soient proportionnées

que ce soit pour protéger l'activité d'associations d'inspiration religieuse, mais n'organisant pas un culte- je pense aux scouts -, ou pour mettre en place des obligations comptables proportionnées aux sommes reçues. Les contraintes pesant sur les associations relevant de la loi de 1905 comme sur celles qui relèvent de la loi de 1901 seront nombreuses et difficiles à mettre en oeuvre.

Le Sénat avait souhaité préserver les spécificités En effet, si le droit local doit évoluer comme celui du reste de la France, ses spécificités demeurent, puisqu'il n'est pas envisagé de revenir sur le régime concordataire ni sur le statut des établissements publics du culte. Ici encore, nos propositions n'ont pas été retenues et l'alignement du droit local sur le droit national bouleversera sans nécessité des pratiques ancrées et profondément républicaines.

sur lesquels nous avons pu mener avec l'Assemblée nationale un travail constructif qui a abouti à des mesures protectrices et efficaces. Je relèverai simplement qu'il s'agit de dispositions qui, discutées à l'occasion de l'examen de textes antérieurs, ont pu être enrichies de ces travaux et ajustées au regard des décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Finalement, madame la ministre, ce qui nous a le plus manqué pour parvenir à un accord, c'est le temps. Nous partageons le constat du défi auquel nous faisons face

qui imposent de toucher à des libertés constitutionnellement protégées comme la liberté d'association et la liberté de culte, méritaient que le Parlement puisse débattre pleinement, sinon sereinement, des dispositifs envisagés, au travers de deux lectures. accélérée demandée sur ce texte, que rien ne justifiait, n'a fait qu'accentuer les divergences. L'Assemblée nationale, tout aussi soucieuse de ne pas aborder certains sujets que de ne pas se faire rattraper par une actualité qui prouve la difficulté de déterminer le périmètre et les modalités d'application de la laïcité, n'a pas souhaité s'engager sur la voie d'une solution de compromis. C'est donc à regret, face au constat de l'absence de volonté d'un vrai travail commun, que nous proposerons au Sénat d'adopter la motion tendant à opposer à ce projet de loi

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nul besoin de vous rappeler l'attachement du groupe du RDSE aux principes républicains, à la loi de 1905 et, plus globalement, à la laïcité. Ce sont, pour beaucoup d'entre nous, les fondements de notre engagement. Nous y voyons une source intarissable d'émancipation, de liberté, d'égalité et de fraternité. apparaît-elle comme le bras armé de la pensée universaliste, hélas aujourd'hui malmenée par des séparatistes de tous bords qui n'ont que les différences, la couleur et la religion en tête, avec un seul but : diviser, fracturer et détruire un idéal hérité des Lumières. Dire cela nous oblige également à interroger ce modèle, à en corriger les failles, notamment celles d'un ascenseur social en panne, d'une méritocratie à l'arrêt, d'une perte de confiance dans les institutions. Voilà un débat que nous n'avons peut-être pas suffisamment eu et un sujet sur lequel ce projet de loi n'apporte une réponse que trop partielle. Pour en revenir au texte, les dispositions permettant l'élargissement du principe de neutralité dans les services publics ont directement rencontré notre approbation. C'est, à nos yeux, une étape importante qui est franchie, il convient de le souligner. Je regretterai néanmoins que nombre des dispositions dont nous avions permis l'adoption aient été supprimées par l'Assemblée nationale. Je pense à l'obligation pour les directeurs d'écoles privées hors contrat d'être présents effectivement sur le site de l'établissement et pour les professeurs d'être titulaires d'une charge d'enseignement, disposition portée par notre collègue Nathalie Delattre. Il s'agissait là d'une véritable mesure de vigilance vis-à-vis d'établissements dont le nombre croît sans cesse sans que l'on puisse suffisamment les contrôler. Je pense encore à l'amendement de notre collègue Jean-Yves Roux, proposait d'inclure, dans le projet territorial d'éducation, la valorisation de la charte de la laïcité et du principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Notre groupe était plus partagé sur les dispositions concernant l'instruction en famille et le port des signes religieux ostentatoires pour les accompagnateurs scolaires. Certains d'entre nous étaient favorables au régime de déclaration plutôt qu'au régime d'autorisation, estimant que ce dernier viendrait pénaliser une grande partie des familles qui pratiquent l'instruction en famille dans le respect des règles et des programmes. Par ailleurs, ailleurs, nous étions en grande partie favorables à l'interdiction des signes religieux ostentatoires pour les parents accompagnateurs scolaires, considérant qu'ils devaient s'astreindre à la même neutralité religieuse que les enseignants. Globalement, si nous étions en phase avec la majorité sénatoriale sur ces deux lignes, nous étions également une majorité à nous être opposés à la version du Sénat, qui avait franchi une limite en envisageant la suspension des allocations familiales et de rentrée scolaire pour les familles en cas d'absentéisme.

Je le redis, la République par les actes l'emportera toujours sur la République incantatoire. Attachons-nous à la garantir davantage, en luttant contre la fracture territoriale, en ravivant l'égalité des chances pour que, de nouveau, ce projet commun de République ait un sens.

vampirisé par toute une série d'amendements stigmatisants, visant à interdire les signes religieux aux accompagnatrices scolaires ou à l'université ou encore à interdire le burkini.

Aussi, plutôt que de débattre du séparatisme social, qui gangrène le vivre ensemble dans notre pays, la majorité sénatoriale a préféré l'alimenter avec des mesures phares de son programme électoral, telles que la suspension des allocations familiales en cas d'absence scolaire.

Si la droite sénatoriale a eu le loisir de mettre en débat et de faire adopter ses mesures d'exclusion parfois discriminatoires dans un élan de surenchère sécuritaire porteur d'amalgames, c'est que le Gouvernement l'y a invitée en présentant un texte aux antipodes des objectifs qui lui avaient Car, mes chers collègues, qui ne veut pas renforcer les principes de notre République ? Personne ! Mais la définition de ces principes et de ce qu'ils renferment est-elle univoque ? Fait-elle consensus ? Loin de là Selon nous, les principes de la République- ses valeurs -sont notre bien commun, car ils déclinent ce qui devrait assurer que personne ne soit oublié par elle. Alors que, selon nous, laïcité rime avec progrès social et liberté de conscience, c'est en s'appuyant sur une tout autre définition de la laïcité que le Gouvernement justifie à l'inverse des mesures de contrôle et d'ordre public. Une vraie lutte contre l'islamisme politique, si l'on avait vraiment voulu ouvrir le débat, aurait nécessité que l'on se penche aussi sur nos relations internationales de complicité avec de nombreux États dans le monde qui organisent l'islamisme politique et oppriment leur propre population, souvent musulmane. L'erreur de la droite en se positionnant ainsi a été de permettre au Gouvernement d'apparaître comme plus soucieux des libertés publiques, alors que nombre des dispositions de son texte initial étaient déjà très attentatoires à ces telles que la tutelle sur les associations ou le régime d'autorisation auquel seront désormais soumis les cultes, ce texte néoconcordataire est marqueur d'un recul sans précédent sur la loi de 1905, de 1905, laquelle avait été élaborée par un législateur ayant les idées claires, comme le souligne l'historien et politologue Patrick Weil- je le cite : « En séparant les Églises et l'État, il voulait rompre avec le régime de l'administration par l'État des cultes. » ce texte porte atteinte, par petites touches, aux équilibres de la loi de 1905, aux libertés de culte, d'association et d'enseignement, recelant controverses et crispations. Nous exprimons de nouveau, aujourd'hui, notre opposition à cette vision,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici à nouveau réunis, après des heures de débat dans cet hémicycle, pour discuter de ce projet de loi, dont l'objet affiché était, paraît-il, de conforter les principes de la République.

Une promesse de cohésion autour de valeurs communes. Une promesse d'émancipation pour chacun, indépendamment des conditions de départ dans la vie. Une promesse de justice sociale et de solidarité. La République, c'est le ciment de notre société, autour des trois mots qui la célèbrent : liberté, égalité, fraternité. En octobre, Emmanuel Macron soutenait que « la République c'est à la fois un ordre et une promesse ». S'il y a bien des mesures d'ordre dans le présent projet de loi, où est passée la promesse ? Plus d'un tiers des articles instaurent des procédures de contrôle, plus d'un quart définissent des peines d'emprisonnement. Plus grave, certaines dispositions sont dangereuses, pour nos libertés et celles de nos concitoyens. C'est le cas, bien sûr, de l'article 18, mais aussi de l'ouverture d'une possibilité de recours à la comparution immédiate pour les contentieux des abus de la liberté d'expression. Écologiste et Républicain n'acceptera jamais de rogner sur nos libertés pour une chimère de sécurité. L'ordre donc. Mais où est la promesse ? Pas un mot sur la mixité sociale, la lutte contre les discriminations, l'éducation populaire, l'accès aux services publics. Comment défendre les principes de la République, si l'on ne s'attache pas à en faire respecter les valeurs ? Comment défendre la République, si l'on ne s'assure pas que ses promesses sont les mêmes pour tous sur notre territoire, que ce soit en matière de logement, d'éducation ou de santé ? Les élus- ceux que nous sommes comme les élus locaux -savent pertinemment que, sans traitement de ces sujets, le texte est infirme. Notre groupe ne s'est pas opposé à toutes les mesures du projet Nous sommes toujours favorables au renforcement de la protection des agents du service public et, bien évidemment, à toutes les dispositions visant à lutter contre les pratiques portant atteinte à la dignité des femmes. Nous n'éludons pas la nécessité de combattre l'islamisme radical et la radicalisation. Nous l'avons fait à plusieurs reprises sans faillir. Nous ne sommes pas aveugles aux difficultés, mais nous considérons que cette lutte ne saurait passer par une stigmatisation à outrance de citoyens français en raison de leur religion. Ce texte restera avant tout un texte de défiance : envers les croyants, envers les bénévoles des associations, envers l'école et, au fond, envers tous les citoyens. Après l'échec de la commission mixte paritaire, nous ne pouvons qu'être satisfaits de la suppression par l'Assemblée nationale des dispositions iniques votées par la majorité du Sénat. Je pense, bien évidemment, à l'interdiction d'accompagnement des sorties scolaires pour les mères voilées, l'interdiction des drapeaux dans les cérémonies de mariage, à la suppression des allocations familiales en cas d'absences d'un élève ou encore aux mesures sur l'instruction en famille. Ainsi, la droite sénatoriale a réussi le tour de force de permettre au Gouvernement d'apparaître comme modéré sur ce sujet. C'est un comble

Nos propositions existent toujours. Nous sommes prêts à les défendre à nouveau dans cet hémicycle, car nous considérons que le texte revenu de l'Assemblée nationale n'est toujours pas à la hauteur. Nous regrettons ainsi que nos collègues députés aient supprimé les dispositions visant à faire respecter la laïcité, par exemple sur le matériel électoral. Nous proposons de les réintroduire. La protection de la liberté d'association, un des fondements de la République, est au coeur des valeurs de gauche. Les dispositions de l'article 6, conditionnant l'octroi de subvention à la signature d'un contrat d'engagement républicain, sont non seulement inutiles, mais dangereuses. Elles placeront les associations dans une insécurité et instaurent un climat de suspicion, alors que de nombreuses associations pallient les déficiences de l'État sur des pans entiers de notre territoire national. Nous en proposons donc la suppression. Parce que la défense des droits des femmes est essentielle à nos yeux, nous présentons plusieurs amendements visant à la renforcer, notamment s'agissant des certificats de virginité. Notre groupe a également à coeur de défendre la liberté de la presse. C'est l'objectif de l'amendement que nous avons déposé pour modifier l'article 18, et ce afin de garantir que ses dispositions ne nuisent ni à la liberté d'expression ni à celle d'informer. D'autres amendements, enfin, concernent les dispositions relatives aux associations cultuelles. Nous n'oublions pas que c'est la République qui assure la liberté de pensée, de conscience et de religion, qui garantit la liberté de manifester son appartenance religieuse, comme son absence. C'est le coeur de la loi de 1905 : par la séparation des Églises et de l'État, celle-ci garantit la liberté de chacun, en offrant un cadre commun à tous. Les nouvelles contraintes imposées aux associations cultuelles sont, à cet égard, inquiétantes.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues,

L'islamisme utilise quatre voies d'intrusion : celle de l'immigration et de la démographie ; celle de la dissimulation, ou silencieuse ; celle de la provocation et victimisation ; celle du terrorisme sanglant. Aucune de ces voies n'est prise à bras le corps dans ce texte. Et pour cause ! Le Gouvernement s'est trompé sur la nature de l'ennemi : nous sommes, non pas face à un communautarisme séparatiste, mais face à un communautarisme de conquête soutenu par des idiots utiles de tous bords. Pourtant, l'actualité a tout d'une alerte islamiste supplémentaire qu'on se refuse d'entendre : le 6 juillet dernier, 169 enfants de djihadistes ont été rapatriés en France. Personne pour en parler Quand on connaît la violence des « lionceaux du Califat », enfants soldats de l'État islamique, il est vital que ces enfants soient fichés et surveillés de très près. Au lieu de cela, M. Dupond-Moretti a opposé à cette proposition de votre serviteur, « l'inhumanité » de son auteur. Le garde des sceaux a moins de scrupules, quand il s'agit de ficher les enfants de 12 ans qui ne sont pas vaccinés ou les mineurs en lien avec une personnalité ayant un engagement politique, syndical ou religieux, tel que permis par un décret de M. Darmanin. Par ailleurs, le danger vient de l'extérieur. La résurgence de l'État islamique, le renforcement des groupes armés dans la bande sahélo-saharienne et la montée en puissance des talibans en Afghanistan font peser de lourdes menaces sur notre pays. L'islamisme a le vent en poupe à l'extérieur de nos frontières, comme à l'intérieur. Ce matin même, l'Institut musulman des Bleuets a transformé le parc Chanot, à Marseille, en mosquée géante pour l'Aïd organisation est à l'origine de prêches et de publications islamistes connus du préfet et reconnus par le ministère de l'intérieur. Il semble que la liberté de certains soit devenue sacrée En entame de cette nouvelle lecture, je vous pose la question, mes chers collègues, madame la ministre, combien de Bataclan, de Charlie Hebdo, de promenade des Anglais, de Laura et Mauranne, de père Hamel, d'écoles Ozar Hatorah ? Combien d'Arnaud Beltrame ? Combien de policiers, de professeurs, de militaires français égorgés, décapités ? Combien d'abominations faudra-t-il pour que vous preniez toutes les mesures nécessaires à l'éradication de la lèpre islamiste

le projet de loi que nous examinons s'inscrit dans la lignée de la loi de 1905, texte majeur qui structure depuis plus d'un siècle les relations entre l'État et les religions dans notre pays. La place respective de ces institutions est délimitée par deux repères principaux : la liberté de conscience et la laïcité. Le Gouvernement a souhaité mettre à jour ces dispositions et en ajouter de nouvelles. Les évolutions de notre société ont effectivement rendu nécessaire la précision du cadre civique. Il n'est pas envisageable que des organisations religieuses exercent une quelconque activité politique sur le territoire national, au détriment de notre système démocratique et de nos valeurs républicaines. À cet égard, il nous paraît particulièrement important d'assurer le contrôle nécessaire des financements étrangers dont ces organisations religieuses pourraient bénéficier. bénéficier. Les États étrangers ne doivent pas pouvoir les utiliser comme intermédiaires pour étendre leur influence dans notre pays. Le projet de loi contient d'autres mesures allant dans le bon sens, comme celles qui visent à renforcer la neutralité des agents du service public. Après un examen sérieux et approfondi en première lecture, nous ne pouvons que déplorer l'échec de la commission mixte paritaire dans la recherche d'un texte commun et équilibré. Nous nous félicitons que nos collègues députés aient conservé plusieurs améliorations apportées au texte par le Sénat. Néanmoins, dans sa globalité, la version adoptée en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale ne laisse pas apparaître un esprit de compromis. C'est d'autant plus regrettable que les deux chambres visent les mêmes objectifs.

ce nouveau régime risquait surtout d'être contreproductif et qu'il portait atteinte à la liberté d'enseignement. L'Assemblée nationale a néanmoins décidé de le rétablir, ce que nous regrettons. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la haine en ligne, notre groupe avait déposé un amendement visant à responsabiliser les plateformes. Défendue par le président de notre groupe, Claude Malhuret, et soutenue par notre assemblée, cette disposition de bon sens a été purement et simplement supprimée par la rapporteure Laetitia Avia sur la base d'un argumentaire qui tient plus du tweet que de la démonstration ... Vu l'urgence à agir contre la haine en ligne, il est regrettable que Mme Avia, sur ce sujet a été censurée par le Conseil constitutionnel, s'oppose ainsi aux initiatives tendant pourtant à atteindre le même objectif. Constatant les écarts entre les versions de l'Assemblée nationale et du Sénat, la commission des lois nous propose de voter une motion tendant à opposer la question préalable.

qui avait, en première lecture, motivé un vote contre du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires. Les rapporteures de la commission des lois ont fait le choix de déposer une motion tendant à opposer la question préalable au présent projet de loi, estimant que la majorité La République En Marche à l'Assemblée nationale n'entendait pas « trouver avec le Sénat le moyen de progresser sur les sujets graves que sont la neutralité de l'État, la laïcité et le vivre ensemble, sur lesquels le Sénat avait fait des propositions concrètes en première lecture Je le rappelle, notre groupe avait estimé que ni le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale ni le texte issu des débats au Sénat n'étaient satisfaisants. L'un comme l'autre ne constituent en rien une protection des droits et libertés des Français face aux montées de l'islam radical ; au contraire, ils font courir de nombreux risques d'atteintes à diverses libertés individuelles et fondamentales, telles que la liberté de culte, la liberté de conscience ou la liberté d'association. Nous voterons également contre la motion déposée par la mais nous tenons à réaffirmer notre opposition au présent texte, qui n'est que la conséquence de l'échec des politiques d'intégration, d'égalité et de cohésion sociale menées par les gouvernements successifs depuis des années. L'inégalité sociale dans notre pays est l'un des véritables séparatismes majeurs. Selon l'Observatoire des inégalités, tous les indicateurs montrent une progression des inégalités en France. Pour exemple, 30 % des élèves de l'École polytechnique sont issus de seulement deux lycées parisiens. Pendant ce temps, les élèves des banlieues ou des territoires ruraux sont les principaux décrocheurs du système scolaire. Une vraie réforme de fond sur les facteurs de clivages sociaux aurait ainsi mieux permis de redonner l'envie de faire société. Face aux faux débats qui appauvrissent la pensée, nous nous devons de rappeler notre profond attachement à la laïcité et à la liberté de conscience, telles qu'elles sont inscrites à l'article 1 de la loi de 1905. Celle-ci donne le droit de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion ; elle donne finalement le droit à l'indifférence bienveillante de notre République. La laïcité ne peut en aucun cas être utilisée pour stigmatiser et exclure une partie de nos concitoyens de la communauté nationale. Ce projet de loi, assorti de contrôles, de répressions et d'interdictions visant les associations cultuelles, constitue un empiétement du politique sur le religieux. Quand le religieux devient politique, il y a danger pour la démocratie, mais inversement le politique ne doit pas se mêler de religieux. Le renforcement du pouvoir de contrôle de l'autorité administrative, aux dépens de l'autorité judiciaire, déstabilisera à court terme l'équilibre de la séparation entre églises et État. En outre, l'État dispose d'ores et déjà de moyens juridiques pour lutter contre les dérives sectaires et l'apologie de la violence, même s'il peine à faire appliquer la loi. Plutôt qu'une production pavlovienne de mesures réactionnaires, il aurait été opportun d'octroyer les moyens nécessaires à cette lutte, là où sévissent ces dérives. À l'aune des crises qui s'enchaînent et s'entremêlent, monopoliser notre temps législatif avec une succession de textes toujours plus sécuritaires, toujours plus liberticides et ne se penchant jamais sur les réelles causes des vrais séparatismes qu'ils entendent traiter est regrettable.

Il aurait pu être un texte de notre commission, aussi, en cohérence avec le diagnostic majoritairement partagé sur nos travées de la nécessité de se doter des outils juridiques pour répondre à la dynamique de fragmentation exercée par les lois particulières sur la norme commune. La commission des lois a toutefois fait un choix différent, en adoptant une motion de ses rapporteures, ce qui nous conduit, aujourd'hui, à examiner le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Certes, nous ne le déplorons pas sur le fond, car cette version nous semble intégrer des dispositions utiles et équilibrées pour concourir à l'objectif de conforter les principes de notre République. Je pense aux articles relatifs au service public, avec notamment le nouveau délit de séparatisme, au contrat d'engagement républicain qui donnera une assise légale aux décisions des élus locaux, au renforcement de la lutte contre la haine en ligne en cohérence avec la dynamique européenne. à certaines mesures techniques particulièrement bienvenues visant la transparence des financements étrangers et l'incitation des associations à rejoindre le régime de la loi de 1905 pour leurs activités cultuelles, afin de permettre un meilleur contrôle de l'utilisation des subventions publiques. Sur tous ces points, on a d'ailleurs pu constater, dès la première lecture, une convergence entre les deux assemblées. Les modifications apportées par le Sénat sur ces sujets, si elles n'ont pas toutes été conservées lors de l'examen à l'Assemblée nationale

Il nous ramène en fait à l'un des principaux points de désaccord ayant conduit à l'échec de la commission mixte paritaire : l'extension, par la majorité du Sénat, du champ d'application de l'obligation de neutralité et de l'interdiction du port des signes religieux dans l'espace public. Le choix de poursuivre le travail en nouvelle lecture aurait certes exposé la majorité sénatoriale au risque d'un nouveau rejet en commission, comme en première lecture, de ces dispositions relatives à l'interdiction des signes ostensibles. Mais, dans le même temps, ce parti pris audacieux aurait permis d'approfondir un débat sur des mesures dont la majorité reconnaît l'utilité. Nous regrettons donc vivement le rejet du texte qui donne, au détriment d'un examen approfondi de dispositions sur lesquelles nous sommes en mesure de nous accorder, la priorité à des mesures faisant à notre sens dévier le projet de loi de son objet et le fragilisant juridiquement. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe RDPI soutient le texte, tel qui nous arrive de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Ses mesures sur la neutralité du service public, l'école républicaine, la lutte contre la haine en ligne, la protection de la dignité de la personne humaine ou encore le contrôle des financements s'inscrivent dans la continuité de l'esprit libéral de la loi de séparation, dans le respect de sa conception du principe de laïcité- une acception qui implique la neutralité de l'État et la liberté de conscience, non le silence des opinions religieuses de chacun ou l'éviction du religieux de l'espace public.

Dans ce cadre, les deux organismes perçoivent des fonds en provenance de puissances étrangères- cela tombe bien, c'est ce que l'on voulait éviter ! Le montant total des financements étrangers est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. L'importance des financements étrangers, ainsi que le manque de transparence de la part de l'association et du fonds de dotation,

pourquoi ne pas lui donner les moyens législatifs d'assurer sa mission ? L'Assemblée nationale a également supprimé des dispositions de l'article 30 qui prévoyaient que tout projet de construction d'un lieu de culte par une association cultuelle devait être soumis à l'élaboration d'un plan de financement prévisionnel mentionnant l'origine des fonds, certifiée

Malheureusement, le projet de loi sur le séparatisme est devenu « projet de loi confortant le respect des principes de la République » et, au fur et à mesure que le titre s'affadissait,

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances

la citoyenneté prime toute appartenance, entre autres religieuse. La France croit en la République émancipatrice.

cette motion a pour objet d'opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, confortant le respect des principes de la République. En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a supprimé

l'article 18, la volonté du Sénat de poser des distinctions claires permettant le respect par tous des principes de la République, tout en préservant la liberté de culte, n'a pas été entendue.

aucun des mécanismes adoptés par notre assemblée en première lecture qui visaient à préserver le rôle des associations d'inspiration religieuse, sans organiser l'exercice d'un culte, et à simplifier les démarches des petites associations établies de longue date. Par ailleurs,

de parvenir à un texte commun. La présente motion tire les conséquences de cette impossibilité, que nous pouvons tous regretter.

que cette procédure doit être réservée à des circonstances exceptionnelles. Or elle est devenue banale. Cela signifie que nous renonçons au travail que certains et certaines d'entre nous ont connu dans des temps passés,